groupe socialiste et républicain, de la proposition de loi visant à proroger l'expérimentation de la tarification sociale de l'eau prévue à l'article 28

Comme le souligne le Comité national de l'eau dans son rapport de 2017, « sans prolongement de l'expérimentation, légalement engagée pour une durée de cinq ans, les délais de mise en oeuvre des projets font que les collectivités ne disposeront au mieux que de trois ans de recul pour évaluer l'efficacité et l'efficience de leur dispositif, la plupart ne disposant que d'une ou deux années pour expérimenter leur dispositif ». Ce texte répond par conséquent à une demande forte des collectivités et des groupements engagés dans l'expérimentation.

prévoyant l'accès de toutes les personnes physiques à l'eau potable pour leurs besoins essentiels dans des conditions économiquement acceptables par tous. L'accès à l'eau potable reste un enjeu de grande ampleur. Vous le rappelez dans votre rapport, Au total, parmi les 50 collectivités et groupements qui ont été retenus par deux décrets successifs en avril et juillet 2015, quelque 47 se sont effectivement engagés dans l'expérimentation- 38 en métropole et 9 outre-mer. En avril 2017, soit un an avant l'échéance fixée par la loi Brottes, seulement la moitié des projets étaient mis en oeuvre. Ce décalage s'explique par le temps nécessaire à l'État pour mettre en place le cadre général de l'expérimentation, mais également par le temps nécessaire aux collectivités, qui présentent d'un point de vue démographique et statutaire des profils très variés, pour déterminer les solutions les plus adaptées : quelles seront les populations bénéficiaires, et selon quels critères ? Quels interlocuteurs retenir pour la mise en oeuvre ? Quel dispositif d'aide sera le plus adapté à la spécificité des territoires selon, par exemple, la part d'habitat individuel et collectif ? À combien s'élèveront les coûts de gestion selon le cadre retenu et au regard du volume d'aide apporté ?

Parce qu'il permet de sécuriser, de reconnaître et de respecter l'engagement de nos élus, afin de faciliter l'accès à l'eau des plus modestes, je me réjouis que la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, sur la base du rapport de Françoise Cartron, dont je salue le travail, se soit prononcée en faveur de ce texte à la quasi-unanimité. J'espère que, toutes et tous, nous suivrons cette position, parce que nous sommes toutes et tous convaincus que ce bien fondamental qu'est l'eau et la problématique de la précarité hydrique seront au coeur de nos débats dans les décennies à venir.

je n'en doute pas, de la nécessité de permettre à nos collectivités locales de poursuivre cette expérimentation pour honorer leurs engagements et tirer les enseignements nécessaires à la mise en place de dispositifs qui soient viables, pérennes et efficaces. Notre position n'est pas isolée ; elle est partagée par le Conseil national de l'eau et par le Conseil général de l'environnement et du développement durable, qui, dans un rapport de février 2016, préconisait de conforter, voire d'accélérer l'expérimentation permise par la loi et de la coordonner avec le dispositif du chèque énergie. La proposition de loi que je défends avec Monique Lubin, Patrick Kanner et le groupe socialiste a été votée par la commission, et je formule simplement le souhait qu'elle connaisse le même sort aujourd'hui en séance publique. À ce titre, je tiens à remercier personnellement Françoise Cartron de la qualité de son rapport et des amendements proposés par la commission, qui vont, me semble-t-il, dans le bon sens. La présente proposition de loi appelle deux réflexions. La première porte sur le droit à l'eau et le service public. Ainsi que l'a rappelé ma collègue Monique Lubin, l'expérimentation de la tarification sociale de l'eau permet d'identifier des solutions adaptées pour une traduction concrète du droit à l'eau, dont je rappelle qu'il est inscrit depuis 2006 dans le code de l'environnement. Je rappelle également que l'Assemblée générale des Nations unies, au vu de l'enjeu géopolitique qu'elle représente, reconnaît l'eau comme un bien essentiel de l'humanité. Notre code de l'environnement dispose pour sa part que « l'eau fait partie du patrimoine commun de la Nation », et que chacun « a le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous ». Comme vous le savez sans doute, les questions du droit et de l'accès à l'eau font partie de l'ADN du département des Landes.

Il pensait en effet que « notre société doit garantir à tous un accès à l'eau potable et à l'assainissement. L'eau n'est pas une marchandise, c'est un bien commun qu'il convient de préserver. » mais l'intervention de la puissance publique demeure pertinente pour faire respecter un droit d'accès à l'eau pour tous, ce à quoi peut justement contribuer l'expérimentation dont nous débattons aujourd'hui.

L'expérimentation de la tarification sociale de l'eau a été rendue possible par l'autorisation accordée aux collectivités locales de déroger, à titre expérimental, aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur,

de l'égalité et de l'intérêt général. Je tiens d'ailleurs à saluer l'ensemble des collectivités qui se sont lancées dans cette expérimentation pour l'adapter au plus près de leur réalité locale. Il faut saluer le courage politique des élus et la mise en musique ingénieuse de leurs services administratifs.

que les territoires sont capables d'innover, de trouver des solutions adaptées à la diversité pour mener des politiques publiques ayant du sens pour nos concitoyens, singulièrement, en l'espèce, pour les plus fragiles d'entre eux. Elles font la démonstration que les territoires ne sont pas un problème, mais une solution, à la condition qu'une relation de confiance existe, que les moyens nécessaires à la libre administration demeurent et que cette dernière serve utilement et équitablement les territoires comme les citoyens. Aussi, pour toutes ces raisons- trouver des solutions adaptées à la concrétisation d'un droit fondamental reconnu internationalement, permettre que les efforts déployés par nos collectivités portent leurs fruits et faire confiance aux territoires -, nous vous invitons, mes chers collègues, à voter pour cette proposition de loi.

Madame la présidente, monsieur le ministre d'État, mes chers collègues, en 2006, le législateur a inscrit dans le code de l'environnement le principe d'un droit à l'eau potable, afin de permettre à l'ensemble de la population d'accéder à l'eau pour ses besoins essentiels dans des conditions économiquement acceptables pour tous. En effet, l'accès à l'eau constitue toujours un sujet essentiel dans notre société. Selon un rapport du Conseil général de l'environnement et du développement durable de 2011, la facture d'eau et d'assainissement dépasserait le seuil d'acceptabilité, fixé à 3 % du revenu, pour près de deux millions de Français. Face à une telle situation, de nombreux élus locaux, toutes sensibilités politiques confondues, ont engagé depuis plusieurs années des actions en faveur d'une véritable politique sociale de l'eau. Afin d'encourager et de sécuriser ces initiatives, la loi du 15 avril 2013, également appelée « loi Brottes », permet aux collectivités territoriales qui le souhaitent de s'engager dans une expérimentation en application de l'article 72 de la Constitution, les autorisant à déroger à titre expérimental et pour un objet et une durée limitée aux dispositions qui régissent l'exercice de leurs compétences. L'expérimentation, créée en 2013, donne ainsi la possibilité aux collectivités et à leurs groupements de tester différents dispositifs sociaux, afin de faciliter l'accès à l'eau des ménages les plus modestes. Concrètement, elle permet aux collectivités de mettre en oeuvre une tarification sociale de l'eau, de verser des aides aux usagers ou encore d'accroître leur contribution au Fonds de solidarité pour le logement, le FSL, afin de résorber les impayés. Les collectivités volontaires pour participer à l'expérimentation devaient transmettre une demande au préfet de leur département avant le 31 décembre 2014. Au total, cinquante collectivités et groupements ont été retenus. Ces participants présentent des profils très variés en termes de statut, d'importance démographique ou de caractéristiques locales. L'expérimentation fédère ainsi des communes, des EPCI à fiscalité propre, des syndicats mixtes, issues de territoires aussi bien urbains que ruraux, dont certains se caractérisent par une part importante de logements locatifs, tandis que d'autres accueillent un nombre élevé de résidences secondaires.

Toutefois, comme le rappelle un rapport d'étape du Comité national de l'eau publié en 2017, l'expérimentation a fait l'objet d'une mise en oeuvre très progressive. Ainsi, en avril 2017, soit un an avant l'échéance fixée par la loi Brottes, seulement la moitié des projets étaient mis en oeuvre. Ce décalage s'explique par le temps nécessaire à la fois pour que l'État puisse mettre en place le cadre général de l'expérimentation et pour que chaque collectivité puisse définir et déployer les solutions les plus adaptées au contexte local. Sans prorogation, les collectivités ne disposeront au mieux que de trois années de recul, et pour la plupart d'entre elles de seulement un à deux ans de mise en oeuvre effective. L'ensemble des parties prenantes considère que cette durée est trop brève pour évaluer pleinement les effets de l'expérimentation. Les premiers résultats sont toutefois prometteurs et riches d'enseignements. les collectivités participantes ont conçu des solutions innovantes et diversifiées en tenant compte des spécificités locales. La modulation tarifaire a été retenue lorsque les abonnés individuels représentaient une part significative des usagers. Certains territoires ont ainsi choisi de mettre en place une tarification à la fois environnementale et sociale, conjuguant une approche solidaire et pédagogique quant à la préservation de la ressource. Pour l'habitat collectif, dont les usagers ne sont pas abonnés directement au service d'eau potable, les collectivités privilégient des aides préventives, afin de permettre aux foyers modestes de régler tout ou partie de leurs dépenses liées à l'eau, ou un financement accru au FSL et aux centres communaux d'action sociale pour résoudre les situations d'impayés. Sur plusieurs points, les données et les retours d'expérience doivent être encore consolidés. Il s'agit notamment du coût de gestion des différents dispositifs, de l'évolution du nombre d'impayés et de l'évaluation de l'effet de ces aides sur la consommation d'eau. Cette expérimentation très intéressante mérite donc d'être prolongée, afin d'en tirer des enseignements suffisamment fiables et exhaustifs pour l'avenir de la politique de l'eau. est l'objet de la présente proposition de loi, déposée le 7 février 2018 par nos collègues Monique Lubin, Éric Kerrouche, Patrick Kanner, ainsi que par des membres du groupe socialiste et républicain, qui vise à proroger l'expérimentation jusqu'au 15 avril 2021, soit un délai supplémentaire de trois ans, au bénéfice des collectivités et groupements déjà engagés dans ce processus. Lors de l'examen du texte, notre commission a largement confirmé l'intérêt de cette prorogation. Les collectivités qui sont engagées dans l'expérimentation y sont très favorables.

Notre commission n'a donc apporté que des ajustements au texte initial. Nous avons notamment privilégié une prorogation de droit de l'expérimentation, en supprimant l'obligation pour les collectivités territoriales d'effectuer une nouvelle demande auprès du préfet du département, notre objectif étant de simplifier la poursuite de l'expérimentation pour les élus locaux. Notre commission a également apporté certaines précisions à la loi du 15 avril 2013, notamment sur la transmission des données à caractère social nécessaires à l'identification de la population bénéficiaire des dispositifs proposés. Au regard des premiers retours d'expérience, il semble en effet utile d'harmoniser les relations entre les collectivités et les organismes de sécurité sociale, pour faciliter la poursuite de l'expérimentation. Je précise que, en application de la législation organique, le dépôt de cette proposition de loi a pour effet de prolonger la durée de l'expérimentation jusqu'à son adoption définitive, pour un délai maximum d'un an.

que ce texte puisse être rapidement inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, pour être définitivement adopté dans les meilleurs délais. Permettez-moi de saluer l'engagement des élus locaux, animés d'une volonté politique forte, volonté nécessaire pour la réussite d'une telle démarche expérimentale. Il serait regrettable que l'expérimentation s'interrompe brutalement, sans que tous ces efforts aient pu porter leurs fruits.

montre combien il est utile de mettre à la disposition des collectivités une gamme d'instruments suffisamment étendue qui réponde au mieux aux besoins de la population en tenant compte du contexte local. La solution optimale pour une grande agglomération ne sera pas forcément la plus pertinente pour un territoire rural. Le législateur devra donc tenir compte de cette diversité avant de généraliser certains dispositifs à l'issue de l'expérimentation. Pour conclure, à l'heure où une révision constitutionnelle visant notamment à développer les facultés d'expérimentation est à l'étude, cette expérience témoigne une fois encore des formidables capacités d'innovation qui existent dans nos territoires et qui méritent amplement d'être soutenues. Sachons faire confiance aux intelligences locales, afin de mettre en oeuvre des réponses adaptées aux grands défis qui nous sont posés, tel l'accès à l'eau

les sénateurs, les philosophes de l'Antiquité, quand ils disaient que l'eau est le principe de tout, ne se trompaient pas ! Pour ma part, je suis convaincu que l'eau est aussi le déterminant de tout, et si nous sommes capables, comme vous le proposez, d'additionner nos intelligences et nos volontés pour préserver cette ressource et mieux la partager, la partager, la paix est envisageable au XXIsiècle. À l'inverse, elle ne l'est pas si nous gâchons ce bien vital. Vous l'avez rappelé, l'eau est le substrat de la vie et un patrimoine commun de la Nation.

par le défi démographique, qui, en se combinant au défi climatique, provoquera des tensions sur une ressource essentielle pour nos concitoyens dans leur quotidien, mais également pour notre environnement, pour notre agriculture et pour notre industrie.

Déjà, dans les premières années du XXIsiècle, les signes précurseurs de ces tensions sont devenus palpables. On a connu au cours de l'été 2017 une sécheresse assez inédite et, dans certaines zones urbaines d'Europe, en raison notamment de la faiblesse de l'entretien des réseaux, des pénuries et des coupures ont fait leur retour. Nous n'en sommes pas là, grâce notamment à la robustesse du modèle français de l'eau.

vise ainsi à prolonger l'expérimentation de la tarification sociale de l'eau prévue à l'article 28 de la loi du 15 avril 2013, dite loi Brottes.

L'article 1 de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques affirme par exemple que « l'usage de l'eau appartient à tous et [que] chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous.

Grâce à la loi Brottes du 15 avril 2013, quelque cinquante collectivités de France métropolitaine, mais également d'outre-mer, se sont portées volontaires et ont mis en place, simultanément, de nouvelles tarifications de l'eau et de l'assainissement l'assainissement et des systèmes d'aide au paiement de la facture d'eau, afin de garantir un meilleur accès à ces services pour les plus démunis. Les dispositifs qui ont été mis en place sont variés : ils ont été établis en fonction du contexte local,

En complément, nombre de collectivités territoriales ont également mis en place une démarche de sensibilisation aux économies d'eau, afin d'accompagner la réduction de la dépense des ménages.

de créances. La plupart ont souhaité aller plus loin grâce à l'expérimentation, en mettant en place des dispositifs plus lisibles et une offre positive à l'égard des populations les plus fragiles, sans attendre que les difficultés de la vie ne conduisent ces populations à ne plus payer leurs factures.

elle a conduit les équipes administratives et les élus à s'interroger sur des habitants en grande difficulté, qui tentent par tous les moyens de régler leurs factures, mais se débattent aussi au coeur des précarités multiples que j'ai précédemment évoquées- difficultés de transport,

et réfléchir à une approche globale des foyers provisoirement et parfois, malheureusement, durablement éloignés du confort digne d'un pays comme la France.

s'il est intéressant ou non de généraliser certaines solutions ou d'adapter notre législation en conséquence. Dans ce contexte,

Madame la présidente, monsieur le ministre d'État, monsieur le président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, mes chers collègues,

l'accès de tous à l'eau, patrimoine commun de la Nation, comme M. le ministre d'État l'a souligné, dans des conditions économiques raisonnables, aussi bien pour les usagers que pour les collectivités de loi destinée à proroger l'expérimentation de la tarification sociale de l'eau, censée s'achever le 15 avril prochain, pour les communes déjà engagées dans l'expérimentation. Moins de cinquante collectivités territoriales et groupements ont été identifiés par décret pour y participer. Par principe, mon groupe parlementaire est favorable au recours aux expérimentations dans le cadre de l'article 72 de la Constitution. En effet, s'appuyer sur des territoires pilotes avant la généralisation d'un dispositif est plus sage, tout particulièrement dans un secteur, celui de l'eau, qui relève de nombreux domaines de compétences régaliennes. ailleurs, nous faisons une confiance totale aux élus locaux, qui connaissent parfaitement la complexité de leur territoire, des enjeux et des solutions qu'il faut apporter. Tout ce qui peut encourager la liberté d'action des élus locaux doit donc être valorisé, quand bien même l'expérimentation ne nous semble pas systématiquement indispensable. Dans ce cas précis, d'ailleurs, elle soulève un certain nombre d'interrogations. Tout d'abord, la tarification sociale progressive de l'eau rompt partiellement avec le principe d'égalité de traitement des usagers devant le service public. L'accès à l'eau potable et à l'assainissement est un droit fondamental. Il faut le respecter. Mais il est aussi de notre responsabilité de trouver un mécanisme de solidarité qui ne mette pas à mal le modèle économique de l'eau, notamment en exerçant une forte pression financière sur les collectivités De plus, un certain nombre d'aides qui peuvent être accordées aux ménages en difficulté existent déjà. Je pense à la possibilité d'appliquer une tarification progressive de l'eau pour les immeubles collectifs d'habitation. Je pense aussi à l'aide du Fonds de solidarité pour le logement. Enfin, selon le rapport d'étape élaboré par le Comité national de l'eau, les collectivités territoriales ont autant recours à une approche dite curative, qui existait avant que l'expérimentation ne soit instituée, qu'à une approche dite préventive.

vise à proroger jusqu'au 15 avril 2021 l'expérimentation de la tarification sociale prévue par la loi Brottes au bénéfice des collectivités territoriales et groupements déjà concernés. Je tiens à saluer l'initiative du groupe socialiste et républicain qui nous permet, à travers ce texte, de soutenir la démarche novatrice et solidaire engagée par nos élus locaux et d'évoquer ainsi un sujet éminemment important. L'objectif de cette expérimentation est d'identifier des solutions pour assurer à chacun l'accès à l'eau potable pour ses besoins essentiels, dans des conditions économiquement acceptables pour tous. tous. Il faut le dire, car c'est une réalité : il existe une cruelle contradiction entre le statut naturel et universel de l'eau et son statut économique et social.

C'est au nom de ce principe que le droit d'accès à l'eau potable et à l'assainissement a été inscrit dans le code de l'environnement, en 2006. C'est au nom du même principe que l'expérimentation d'une tarification sociale de l'eau a été autorisée par la loi Brottes. Mais, nous le savons, une loi, c'est aussi beaucoup de patience, lorsqu'il s'agit de relever un défi aussi immense que celui de l'accès à l'eau potable. Notre rapporteur a rappelé les travaux du Conseil général de l'environnement et du développement durable évaluant à deux millions le nombre de Français qui auraient une facture d'eau et d'assainissement supérieure au seuil d'acceptabilité, estimé à 3 % du revenu. J'insisterai encore davantage sur la gravité de la situation en rappelant que la distribution d'eau potable n'est quantitativement plus- ou pas encore -assurée dans plusieurs territoires ultramarins- je regarde notre collègue de Saint-Martin, qui a vécu de très grosses difficultés voilà encore quelques mois. En Guyane et à Mayotte, d'abord, 15 % à 20 % des habitants n'auraient pas accès à l'eau potable. paradoxe ! La couverture par le service est en effet insuffisante, sous le double effet d'un retard d'équipement et d'une démographie galopante qui, d'une part, densifie les écarts et les zones périurbaines et, d'autre part, fait naître de l'habitat informel. À cela s'ajoute en Guyane un véritable fléau : la contamination des eaux par le mercure résultant d'activités d'orpaillage illégal. Elle pose dans des sites isolés un problème majeur de santé publique dans les villages amérindiens Wayanas du Haut-Maroni, plus de 90 % des enfants présentent des taux de mercure supérieurs aux seuils définis par l'Organisation mondiale de la santé ! En Guadeloupe, ensuite, la vétusté du réseau occasionnerait plus de 50 % de pertes d'eau avant même son arrivée au robinet Résultat : près de 9 % de la population, soit environ 35 000 personnes, sont soumis à des « tours d'eau », c'est-à-dire à des coupures hebdomadaires. Enfin, le prix de l'eau et

C'est pour répondre à ces situations qu'un plan d'action pour l'eau a été lancé lors de la conférence environnementale de 2013. L'un des objectifs est justement de développer la tarification sociale, dont il nous est proposé cet après-midi de proroger l'expérimentation. souligné, la mise en oeuvre du dispositif a été progressive : à la date de la publication du rapport intermédiaire du Comité national de l'eau, soit un an avant le terme de l'expérimentation, la moitié des projets étaient mis en place. seule la communauté d'agglomération du Centre Littoral, soit six communes, dotée d'un service d'eau mieux structuré, a pu opérer une refonte de sa tarification par l'instauration d'une progressivité et d'un « chèque eau

Celle-ci permettra de poursuivre le questionnement sur l'équilibre économique des services d'eau potable et d'assainissement des communes, en prenant en compte les réalités de celles-ci. Si ce retard s'explique par différentes raisons, il révèle avant tout le temps et l'ingénierie nécessaires aux collectivités territoriales pour organiser leurs services, définir les solutions les mieux adaptées et déployer effectivement des dispositifs de tarification ou d'aide. le recensement intermédiaire opéré par le Comité national de l'eau le montre bien, chaque territoire a ses caractéristiques propres. Aussi, du versement d'aides à la modulation tarifaire en passant par l'utilisation accrue du Fonds de solidarité pour le logement, le recours aux différentes dérogations varie d'une collectivité à une autre, démontrant la nécessité de pouvoir adapter la loi au contact du terrain. Par ailleurs, il faudra aussi porter une attention particulière à l'évolution de la consommation d'eau et à toutes les initiatives engagées pour favoriser une consommation responsable. Mes chers collègues, cette expérimentation mérite d'être prolongée, si nous souhaitons disposer d'un recul suffisant pour évaluer les dispositifs et envisager, le cas échéant, la généralisation de certains outils.

Madame la présidente, monsieur le ministre d'État, mes chers collègues, nous examinons cet après-midi une proposition de loi dont l'objet est de permettre la prolongation de l'expérimentation prévue par la loi Brottes. Adoptée en 2013, cette loi d'origine parlementaire a permis aux collectivités territoriales volontaires, sur leurs propres deniers, de mettre en place des outils pour favoriser l'accès à l'eau

Nous ne formulons aucune opposition de principe à cette poursuite, puisque nous avions soutenu, à l'époque, ce dispositif. Pour autant, il faut reconnaître qu'il en faudra beaucoup plus pour garantir le droit à l'eau, tel qu'énoncé par l'article 1de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques. Aujourd'hui, ce droit reste purement fictif : en effet, s'il est possible d'aider les ménages en situation d'impayés, aucun dispositif légal ne permet une aide préventive au paiement de la facture d'eau. Pour notre part, nous nous sommes toujours engagés en faveur d'une aide préventive, privilégiant l'instauration d'une allocation en faveur des ménages dont la facture d'eau dépasse 3 % des ressources. Cette allocation devrait être financée soit par les délégataires de service public, soit par une taxe sur l'eau minérale embouteillée, selon les différentes propositions de loi que nous avons présentées ou soutenues. L'une de ces propositions de loi est en cours de navette. Son adoption définitive permettrait, au-delà des expérimentations prévues par la loi Brottes, de disposer d'un mécanisme directement applicable sur l'ensemble du territoire national. Pour le reste, évidemment, nous ne nous opposons pas aux autres formes de tarification sociale, encore moins à la gratuité.

aujourd'hui trop livrées à elles-mêmes en la matière. À ce titre, et pour que la poursuite de cette expérimentation ait du sens, nous souhaiterions disposer de l'ensemble des rapports prévus. particulier, nous demandons solennellement au Gouvernement la remise du rapport d'évaluation et de proposition du Comité national de l'eau. Par ailleurs, selon le code général des collectivités territoriales, un rapport d'évaluation aurait dû être remis par le Gouvernement au Parlement avant l'expiration de la durée fixée par la loi pour l'expérimentation, ce qui n'a pas été fait. Pour aller plus loin, il convient de s'interroger sur l'ensemble des dysfonctionnements dans le secteur de l'eau et sur leurs effets en matière de tarification et de péréquation. Comment comprendre que l'ensemble des dispositifs d'accès à l'eau soient uniquement financés par la puissance publique, donc les contribuables, alors même que les majors de l'eau, délégataires du service public, réalisent des bénéfices indécents ? Nous le savons tous : l'eau vaut de l'or ! Ensuite, comment confier aux collectivités territoriales une mission de service public supplémentaire en matière de tarification, dans un contexte où les finances locales sont très dégradées et l'environnement législatif en perpétuelle évolution ? Plus globalement, nous devrions nous demander sérieusement comment sortir de ce schéma où l'on socialise les pertes et privatise les profits Sur le fond, il faut être clair : ce dispositif de tarification sociale reste un dispositif d'accompagnement social. Or, pour nous, la question est plus vaste : c'est celle de la définition d'un service public de l'eau, national et décentralisé, qui permette, notamment, un soutien logistique et d'ingénierie aux collectivités territoriales pour l'exercice de leurs compétences, dans l'intérêt des usagers. Il est de la responsabilité de l'État de garantir non seulement le droit d'accès à l'eau pour tous, mais également la préservation de la ressource. Or, aujourd'hui, les logiques strictement financières des délégataires conduisent à de grandes pertes du fait d'un réseau en très mauvais état. Nous réaffirmons donc que l'eau ne doit pas être considérée comme une marchandise ni comme une source de profits ! Nous en arrivons à la question qui nous semble centrale : le prix de l'eau. Un chiffre devrait nous faire réfléchir : le prix de l'eau est inférieur de 10 % dans les villes qui sont en régie municipale, donc en gestion publique. Au-delà des tarifications spécifiques, il faut donc s'attacher à créer les conditions d'une « démarchandisation » de ce secteur, afin de garantir enfin le droit à l'eau pour tous, tel que défini à l'article 1 de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques.

transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes, dite loi Brottes. L'article 28 de cette loi prévoit que, en application du quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution, une expérimentation visant à favoriser l'accès à l'eau peut être mise en oeuvre pour une période de cinq ans. Cette expérimentation prendra donc fin le 15 avril L'objectif était d'offrir aux collectivités territoriales et à leurs groupements la possibilité de définir des tarifs sociaux tenant compte de la composition ou des revenus du foyer, ou de prévoir un soutien financier au paiement des factures d'eau, afin de favoriser l'accès à l'eau. Or la mise en place de ce dispositif expérimental a été retardée, compliquée même, pour certaines communes. En effet, les collectivités volontaires ont dû travailler en liaison étroite avec les services sociaux et les départements, ce qui ne se fait pas sans un laps de temps suffisant. l'expérience prouve que les services sociaux sont plus ou moins coopératifs sur le territoire national. Les collectivités territoriales concernées, ainsi que le Comité national de l'eau, réclament le prolongement de l'expérimentation. Pourquoi devrions-nous le leur refuser ? plus, cette prorogation est rendue nécessaire par le manque de recul que nous avons par rapport à l'évaluation de l'expérimentation. Vous n'êtes pas sans savoir, mes chers collègues, que toute expérimentation doit être accompagnée de rapports d'évaluation, afin que l'on puisse juger de la pertinence d'une pérennisation législative du dispositif.

de l'eau et le rapport d'évaluation final qui doit être remis par le Gouvernement au Parlement avant l'expiration de la durée fixée par la loi. Il a pu être allégué que l'expérimentation menée jusqu'ici n'était pas probante, seules quarante-sept communes s'y étant engagées. Cette objection ne nous semble pas pertinente, puisque, comme l'a rappelé notre rapporteur, Françoise Cartron, dont je salue chemin faisant l'excellent travail, ces communes couvrent un bassin de population de 10 millions d'habitants, pour 1,12 million de personnes potentiellement concernées par la tarification sociale de l'eau. Ce

Leur capacité d'innovation doit être à la base de notre travail, ce dernier devant s'inspirer et se nourrir de l'expérience du terrain. Mes chers collègues, vous l'aurez donc compris : nous voterons en faveur de la prorogation du dispositif de la loi Brottes jusqu'au 15 avril 2021. S'appliquant uniquement aux communes volontaires déjà engagées, cette prolongation leur donnera,, les moyens de poursuivre l'expérimentation dans de bonnes conditions. Toutefois, cette prorogation reporte la question que nous aurons à nous poser avant la fin de l'expérimentation quel dispositif pérenne devrons-nous prévoir en matière d'accès à l'eau ? L'objectif visé par la loi Brottes et par cette expérimentation, faciliter l'accès à l'eau, fait singulièrement penser à un texte que nous avons examiné voilà un an. Je pense Je pense à la proposition de loi relative au droit à l'eau potable et à l'assainissement, discutée le mercredi 22 février 2017 au Sénat, qui prévoyait la création d'une allocation forfaitaire permettant aux ménages les plus nécessiteux de s'acquitter de leur facture d'eau. Or ce droit à l'eau, si nécessaire puisse-t-il être, ne doit pas être un poids pour nos collectivités territoriales. La charge de l'accès à l'eau pèse pourtant soit sur le département le Fonds de solidarité pour le lorsque la consommation d'eau est facturée dans les charges du logement, soit sur la commune son centre communal d'action sociale, lorsque la facture d'eau est individualisée. La multiplication des charges pesant sur les collectivités territoriales, sans cesse accrues et jamais, ou rarement, compensées, se ressent au bout du compte dans la qualité du service public. Il est du devoir de notre Haute Assemblée de dire : stop ! Au demeurant, rien ne nous garantit qu'un tel droit à l'eau, concrétisé par une tarification sociale ou une aide pécuniaire, soit de nature à siphonner effectivement les besoins actuels en aide curative. Il s'agit là d'une des interrogations auxquelles l'expérimentation, une fois prorogée, devra répondre. Ainsi donc, s'il est nécessaire de proroger l'expérimentation afin d'avoir un véritable recul et de démontrer empiriquement le bien-fondé ou l'inutilité de cette mesure,

Madame la présidente, monsieur le ministre d'État, monsieur le président de la commission, madame la rapporteur, mes chers collègues, l'article 1 de la Charte de l'environnement, texte de valeur constitutionnelle, garantit à chacun de vivre dans un environnement sain, « équilibré et respectueux de la santé

l'eau. L'eau est une ressource rare et vitale- les hommes le savent depuis toujours ; à l'avenir, elle le sera probablement de plus en plus.

tous, et l'accès à une eau de qualité une ligne d'action de nos services de distribution et de nos politiques. La loi Brottes a eu le mérite de remettre ces questions à l'ordre du jour de nos débats politiques. Je crois que nous pouvons tous nous en réjouir, car il reste beaucoup à faire. Le Parlement a voulu alerter les pouvoirs publics au sujet de nos concitoyens dont les ressources sont insuffisantes pour leur permettre d'accéder à l'eau. Il existait auparavant une possibilité de recours au Fonds de solidarité pour le logement. Même si nombre d'élus locaux l'ont pratiquée,

de la pertinence des dispositifs. Les décrets concernant les villes choisies pour l'expérimentation ont tardé à être publiés. Par ailleurs, le rapport du Comité national de l'eau dresse un simple bilan de mi-parcours. Les données sont donc insuffisantes pour prendre une décision. J'espère que les assises de l'eau

Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la rapporteur, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, le 15 avril prochain, nous arriverons à l'échéance de l'expérimentation prévue dans le cadre de la loi Brottes, promulguée en avril 2013 et qui avait pour objectif de garantir l'accès à l'eau potable et de mettre en oeuvre une tarification sociale de l'eau. Je remercie nos collègues du groupe socialiste et républicain de leur initiative indispensable pour prolonger cette expérimentation importante. Il était plus que temps de légiférer

Face à cette réalité, plusieurs communes ou groupements de communes ont pris leurs responsabilités en expérimentant la tarification sociale de l'eau sur leur territoire. Le dispositif leur permet de définir des tarifs sociaux en tenant compte de la composition ou du revenu des foyers. Les collectivités peuvent également prévoir un soutien financier au paiement des factures d'eau en identifiant

un vrai risque d'empilement des dispositifs, au-delà des difficultés à informer les principaux intéressés. De même, Bordeaux Métropole, qui a aussi développé une approche préventive par l'utilisation du « chèque souligne dans sa note de synthèse que le développement du dispositif reste très lié localement à l'engagement des équipes de travailleurs sociaux. Le travail d'information et de reconnaissance du dispositif se poursuit d'ailleurs encore auprès de ces équipes. Ces constats prouvent qu'il est primordial de faire bénéficier ces collectivités

J'ai eu la tentation- je vous l'avoue, madame la rapporteur -d'utiliser ce texte pour restaurer, par un ensemble d'amendements, la proposition de loi « visant à la mise en oeuvre effective du droit à l'eau potable et à l'assainissement »,

qui se sont engagés dans cette démarche expérimentale. Ainsi, les conditions légales seront réunies pour que les expérimentations actuelles puissent produire tous leurs effets, condition indispensable pour parvenir à une évaluation complète de cette mesure d'efficacité sociale

Cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi Brottes du 15 avril 2013 portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau

en effet à rendre l'eau accessible dans des conditions économiques acceptables pour tous. Élément indispensable à la dignité humaine, l'eau ou, plus précisément, le droit d'accès à l'eau potable est loin d'être une réalité pour tous, tant au-delà de nos frontières que sur l'ensemble de notre territoire. Un million de ménages ont accès à l'eau en payant un prix considéré comme excessif par rapport à leurs revenus. Plus de 100 000 personnes ne bénéficient pas d'un accès direct à l'eau et à l'assainissement : je pense plus précisément aux populations des squats. Il y a là une urgence sociale Une cinquantaine de collectivités territoriales ont choisi d'expérimenter les dispositifs proposés. La lecture du rapport d'étape établi par le Comité national de l'eau permet de constater la variété des dispositifs mis en place par les collectivités, qui ont le choix entre le versement automatique d'aides ou l'instauration d'une modulation tarifaire par la définition de tarifs tenant compte de la composition ou des revenus du foyer et pouvant ainsi inclure une première tranche de consommation gratuite. Cette gratuité avait elle-même été expérimentée à Libourne par le maire de l'époque, Gilbert Mitterrand. La présentation effectuée par les collectivités locales qui ont expérimenté cette tarification sociale de l'eau révèle le souci

avec les organismes gestionnaires comme la CAF ou la CPAM pour la transmission des données individuelles, la nécessité d'un travail de sensibilisation avec les délégataires et les bailleurs sociaux, sans oublier une sensibilisation des consommateurs en faveur d'une utilisation économe de l'eau, ce qui constitue l'un des moyens les plus efficaces pour limiter le poids de la facture d'eau dans les foyers. Les collectivités locales qui se sont lancées dans cette expérimentation cherchent à simplifier les procédures pour accroître l'efficacité des dispositifs.

N'oublions pas, comme le répétait Danièle Mitterrand, que « l'eau, c'est la vie ». Ce droit d'accès à l'eau potable ne saurait être réduit à une aide facultative et expérimentale. Avec mes collègues du groupe socialiste et républicain, je voterai ce texte en vous demandant de poursuivre notre réflexion et notre inlassable combat pour la nécessaire inscription du droit à l'eau dans la Constitution ! D'autres États comme la Slovénie ou le Burkina Faso l'ont fait bien avant nous

2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes.

Pourquoi ce rappel historique ? La raison d'être de cette expérimentation est de favoriser la mise en place d'aides préventives plutôt que de s'évertuer à accumuler les dispositifs par nature et trop souvent curatifs. Comme en témoigne l'instruction du Gouvernement en date du 4 mars 2014 relative à la mise en oeuvre de l'expérimentation, cette tarification sociale de l'eau peut prendre plusieurs formes soit une aide au paiement des factures, qui constitue une aide curative, soit une aide à l'accès à l'eau, qui est une aide préventive. Les collectivités locales ont le choix et peuvent ainsi inclure une première tranche de consommation gratuite ou envisager une autre approche fondée sur un barème reposant lui-même sur les caractéristiques des abonnés. L'idée de cette expérimentation, conformément à la philosophie de l'article 72 de la Constitution,

Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, madame la rapporteur, mes chers collègues, je ne peux qu'appuyer les interventions des collègues Cette proposition de loi déposée par le groupe socialiste et républicain répond à de véritables enjeux sociaux et écologiques, ainsi qu'en matière de développement durable. La prorogation de l'expérimentation est nécessaire et doit permettre une plus grande efficacité des dispositifs mis en oeuvre. Les collectivités locales retenues ont pris du retard. Cela résulte du temps consacré à l'élaboration de leur projet. Il est évident que nous nous devons de laisser ces expérimentations se poursuivre.

Il s'agit bien entendu d'aider ces foyers en difficulté en amont, mais aussi de lutter contre la précarité hydrique. Le droit à l'eau est inscrit dans la loi. Si nous avons la chance de disposer de bons services publics de l'eau et de l'assainissement en France, il est nécessaire de faire progresser le cadre réglementaire pour l'accès à l'eau. Il s'agit d'enclencher tous les leviers pour la mise en oeuvre du droit de l'humain à l'eau potable. Cette tarification sociale s'inscrit dans les objectifs de développement durable, les fameux ODD, qui sont au

l'eau potable va coûter de plus en plus cher, car le coût de l'assainissement va augmenter. En effet, nos ressources en eau- je rappelle qu'il s'agit de moins de 1 % de l'eau disponible sur Terre sont de plus en plus polluées et le coût des traitements pour maintenir une eau potable de qualité ne cesse de s'envoler. Aujourd'hui, en France, la moitié des eaux de surfaces ne sont plus potables. Cette dégradation s'explique par la présence de pesticides, de métaux,

de déchets médicamenteux et autres molécules artificielles non dégradables naturellement. Les trois quarts des nappes phréatiques contiennent des nitrates et la question de la mise en oeuvre de politiques publiques de diminution des pollutions

Je vois dans ces expérimentations une responsabilisation de l'usager. La sensibilisation à l'économie de la ressource en eau est symbolisée par l'exemple du mécanisme « éco-solidaire » mis en place dans le Dunkerquois. L'idée selon laquelle « moins l'on consomme, moins l'eau est chère » a permis une baisse générale de la consommation. de conscience par chacun de son « empreinte eau » et l'adoption d'un comportement responsable sont donc au coeur de la proposition de loi que nous examinons. Dernier point que je souhaite évoquer : l'aspect expérimental de la démarche. Comme le disait Léonard de Vinci : « Détourne-toi des préceptes de ceux qui spéculent sur le monde, mais dont les raisons ne sont pas confirmées par l'expérience. L'expérience ne se trompe jamais, ce sont nos jugements qui se trompent.

Les résultats de ces expérimentations seront donc précieux. Cette proposition de loi est un vecteur ambitieux et audacieux. Il l'est d'abord par sa visée sociale.

l'initiative de nos collègues Monique Lubin, Éric Kerrouche, Patrick Kanner, ainsi que des membres du groupe socialiste et républicain, qui ont déposé cette proposition de loi visant à proroger l'expérimentation de la tarification sociale de l'eau jusqu'au 15 avril 2021.

des finances publiques qui aide les élus et le personnel à percevoir les recettes et à trouver des solutions pour les redevables. Le prix de l'eau est très variable d'une commune

Madame la présidente, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, le 18 janvier 2018 -, l'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi visant à faciliter la sortie de l'indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer. Ce texte, qui vous est aujourd'hui présenté, propose des dispositifs innovants et nécessaires pour apporter des solutions pratiques aux difficultés de règlement des indivisions successorales en outre-mer, difficultés auxquelles le Gouvernement est particulièrement sensible. La proposition de loi est née d'une initiative du groupe Nouvelle Gauche et apparentés à l'Assemblée nationale, plus particulièrement de M. Serge Letchimy, député de la Martinique, qui a souhaité porter cette question devant la représentation nationale. Cette initiative heureuse traduit une préoccupation que partagent tous les élus ultramarins, au palais du Luxembourg comme au palais Bourbon, ainsi naturellement que dans les territoires concernés. La problématique en la matière est en effet bien réelle. Le sujet a été particulièrement bien analysé, notamment dans un rapport extrêmement complet de la délégation sénatoriale à l'outre-mer, en date du 23 juin 2016. Ce travail a été coordonné par M. Thani Mohamed Soilihi, aujourd'hui rapporteur au Sénat de cette proposition de loi, que je salue. Ce rapport constitue, à dire vrai, le travail de référence sur cette question. Votre délégation y avait fait le constat de l'existence d'un état généralisé d'indivision transgénérationnelle, rendant difficile toute utilisation ou disposition de la terre, ce qui constituait dès lors un frein aux investissements économiques ainsi qu'un obstacle à l'accès à l'habitat. Il était observé que cette situation pouvait même aller jusqu'à engendrer des troubles à la paix publique. Ce problème d'indivision endémique se double d'une problématique de reconstitution des titres de propriété, qui sont extrêmement difficiles à établir. le plan du contentieux civil, il a été relevé une multiplication des actions en revendication de propriété, conduisant souvent à la formulation de demandes en partage qui engorgent les tribunaux. Les juridictions sont alors confrontées à des difficultés majeures, liées à l'application des règles de gestion de l'indivision de droit commun fondées sur la règle de l'unanimité ou des deux tiers des droits indivis. Cette réalité est bien identifiée par les pouvoirs publics et, bien entendu, le Gouvernement comprend la volonté forte des parlementaires d'outre-mer d'agir. C'est la raison pour laquelle il a porté un regard attentif et ouvert sur la démarche proposée, en suggérant quelques améliorations au dispositif initial. Je rappellerai en préalable que, dès 2009, la question du titrement des terres a été mise en débat. La création d'un groupement d'intérêt public chargé de rassembler tous les éléments propres à reconstituer les titres de propriété dans les départements d'outre-mer et à Saint-Martin, pour les biens fonciers et immobiliers qui en sont dépourvus, a ainsi été autorisée par la loi du 27 mai 2009 Le dispositif a ensuite été amélioré et complété par la loi du 17 octobre 2013, qui a mis en place une procédure dite de titrement, conduite par un groupement d'intérêt public ayant vocation à être constitué dans chaque région, département ou collectivité d'outre-mer concerné, ou bien par un opérateur public foncier.

possession acquisitive, et les a sécurisés en enfermant les contestations éventuelles dans un délai de cinq ans pour les immeubles situés en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, en Guyane, à Saint-Martin et à Mayotte.

Il est entré en vigueur le 1 janvier 2018. La loi Égalité réelle outre-mer a également créé, pour Mayotte, une commission d'urgence foncière chargée de préfigurer le groupement d'intérêt public. Enfin, en Polynésie française, le tribunal foncier se met en place. Le décret du 16 octobre 2017 relatif à l'organisation et au fonctionnement du tribunal foncier de la Polynésie française est en effet entré en vigueur le 1 décembre 2017. Le Gouvernement convient toutefois qu'il faut aller plus loin sur la question de l'indivision, et ce dans le respect des principes constitutionnels, à savoir le droit de propriété ou le principe d'égalité. C'est dans cet état d'esprit que, dès le dépôt de la proposition de loi, les ministères de la justice et des outre-mer se sont attachés à engager un dialogue constructif avec tous les parlementaires intéressés par ce sujet, naturellement avec l'auteur de la proposition de loi M. Serge Letchimy, mais aussi avec M. Olivier Serva, président de la délégation aux outre-mer à l'Assemblée nationale. Nous avons pu également échanger en amont avec votre rapporteur, pour voir dans quelles conditions ce texte pouvait prospérer. Cette réflexion collaborative a permis une évolution du texte présenté à l'Assemblée nationale. Certaines dispositions demeurant encore perfectibles, le Gouvernement a été particulièrement attentif, lors de la discussion en séance du 18 janvier dernier, à l'amélioration de deux garanties considérées comme essentielles : d'une part, la notification individuelle du projet de partage ou de vente à l'ensemble des indivisaires afin de les mettre en mesure de s'opposer à l'acte et, d'autre part, la saisine du juge par les indivisaires majoritaires en cas d'opposition afin de veiller au respect du droit de propriété de chacun. Les amendements déposés par le Gouvernement sur ces deux points ont été adoptés par l'Assemblée nationale. Il en est ressorti un texte qui me paraît équilibré et solide, tout à la fois porteur de renouveau pour ces successions ultramarines et respectueux des droits en présence. Votre commission des lois a également imprimé sa marque à cette proposition de loi pour en améliorer les termes. Le texte issu de la commission, tel qu'il vous est aujourd'hui présenté, comporte des précisions rédactionnelles supplémentaires, qui me paraissent tout à fait adaptées. Je constate par ailleurs que votre commission des lois a procédé à diverses extensions quant au champ territorial de la proposition de loi, aux fins d'y inclure les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Elle a également prévu d'étendre les dispositions concernant l'attribution préférentielle et l'omission d'héritiers, qui, initialement, ne visaient que la Polynésie française, aux autres collectivités d'outre-mer. Je relève également que le délai pour permettre l'accès au dispositif de vente et de partage a été porté à dix ans, contre cinq ans dans la version adoptée par l'Assemblée nationale, et que le texte étend désormais les pouvoirs de la majorité des indivisaires aux actes d'administration de l'indivision. Le Gouvernement en prend acte et n'entendra pas revenir sur ces modifications, estimées nécessaires par le rapporteur et la commission des lois, dont je salue le président. Seules deux divergences me semblent demeurer à ce stade. Le nouvel article 5 A de la proposition de loi concernant le partage par souche en Polynésie française, adopté sur l'initiative de Mme Lana Tetuanui, renvoie à une question que nous avons déjà évoquée à l'Assemblée nationale avec Mme Maina Sage. C'est un sujet complexe, et je comprends bien entendu les préoccupations des parlementaires de Polynésie. J'ai demandé à mon cabinet et à mes services de mener un travail de fond pour continuer à creuser cette question extrêmement importante. Ce travail a été entamé pendant l'examen de la proposition de loi à l'Assemblée nationale. Il suppose d'y consacrer un peu de temps pour bien mesurer les besoins exprimés et déterminer les réponses juridiques adaptées. Je propose Je propose donc, en lien avec le ministère des outre-mer, que cette réflexion soit conduite de manière plus formelle, avec le soutien de la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice. Je souhaite que les sénateurs et les députés de Polynésie puissent participer à ce travail commun pour trouver les solutions les plus opérationnelles, dans le respect de nos principes fondamentaux. À ce stade, donc, la rédaction de l'article 5 A me semble aller trop loin. Elle ne préserve pas suffisamment les droits de l'ensemble des indivisaires, ainsi que l'accès au juge. Le Gouvernement proposera donc de revenir De même, et c'est le second point de divergence, il sera proposé de revenir sur le nouvel article 2 , qui comporte des dispositions fiscales prolongeant le système d'exonérations fiscales prévu pour Mayotte de 2025 à 2028 et l'étendant aux autres collectivités ultramarines. Au-delà de ces deux points de désaccord provisoire, je me réjouis que nous ayons ici l'occasion, ensemble, de faire évoluer notre droit, avec la perspective de faire progresser de manière concrète la question des successions en outre-mer. Je sais cette considération partagée par ma collègue Annick Girardin, ministre des outre-mer, qui n'a pu être présente aujourd'hui, mais dont l'action est guidée par le souci constant

Madame la présidente, madame la garde des sceaux, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues,

Ce rapport a d'ailleurs largement inspiré la proposition de loi que nous examinons, comme l'ont précisé ses auteurs. Pour une bonne part, les situations d'indivision sont devenues inextricables, car résultant de dévolutions successorales non réglées, parfois même non ouvertes, sur plusieurs générations. Elles stérilisent une grande partie du foncier disponible sur des territoires où celui-ci est rare. L'activité économique, tout comme la politique d'équipement des collectivités en sont entravées. Face à cette situation, nous faisons le constat de règles de gestion de l'indivision inadaptées, en l'état actuel du droit, aux spécificités ultramarines. En application du principe d'identité législative, les départements et régions d'outre-mer sont soumis aux mêmes règles que les territoires hexagonaux, à quelques exceptions près. au décès d'une personne, dans l'attente du partage qui fixera les droits de chacun sur un lot déterminé, les héritiers sont propriétaires indivis des biens du défunt, à moins que celui-ci n'ait réglé les modalités du partage par testament. Cette situation d'indivision n'a pas vocation à perdurer. Selon l'article 815 du code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué [ Toutefois, en application de l'article 815-3 du même code, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte de disposition, tel que la vente ou le partage. Or, en raison du nombre des indivisaires et de leur éparpillement géographique, notamment, l'unanimité est particulièrement difficile à obtenir, ce qui bloque tout projet de vente ou même de réhabilitation des biens. Certes, il existe des procédures spéciales, telles que le partage judiciaire ou la possibilité pour les indivisaires détenant au moins deux tiers des droits indivis de demander au tribunal de grande instance d'autoriser la vente d'immeubles par licitation, mais elles ne permettent pas aux territoires ultramarins de surmonter les difficultés rencontrées. Dès lors, comme les y autorise l'article 73 de la Constitution, les auteurs de la proposition de loi ont souhaité adapter les règles du droit commun aux caractéristiques et contraintes particulières de ces territoires. La proposition de loi, dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, tendait à mettre en place un dispositif dérogatoire et temporaire pour favoriser les sorties d'indivision et encadrer les conséquences des partages qui en découlent. l'article 1, il était prévu que les biens indivis situés dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, et relevant de successions ouvertes depuis plus de cinq ans pouvaient faire l'objet d'un partage ou d'une vente sur l'initiative des indivisaires titulaires en pleine propriété de plus de la moitié des droits indivis. L'article 2 avait pour objet d'autoriser le notaire à accomplir la vente ou le partage à défaut d'opposition des indivisaires minoritaires dans un délai de trois mois suivant la notification du projet. En cas d'opposition d'un ou plusieurs indivisaires minoritaires, les indivisaires majoritaires qui souhaitaient vendre le bien ou procéder à son partage devaient saisir le tribunal. Ce dispositif avait vocation à s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2028. L'article 5, ajouté par l'Assemblée nationale, visait à adapter aux spécificités polynésiennes le dispositif d'attribution préférentielle. On permettrait à un héritier copropriétaire ou au conjoint survivant de demander l'attribution préférentielle du bien, s'il démontre qu'il y avait sa résidence depuis plus de dix ans, alors qu'en application du droit en vigueur, le demandeur doit prouver que sa résidence se trouvait sur le bien « à l'époque du décès » du. L'article 6, également ajouté à l'Assemblée nationale, tendait à empêcher la remise en cause, en Polynésie française seulement, d'un partage judiciaire transcrit ou exécuté par un héritier omis, celui-ci ne pouvant que demander de « recevoir sa part soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage

de propriété. Elle a tout d'abord rappelé que le droit de propriété, garanti par les articles II et XVII de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ne pouvait souffrir de limites à son exercice, à moins que ces limites ne soient justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi. Elle a considéré que la situation tout à fait particulière du foncier ultramarin constituait effectivement un motif d'intérêt général, justifiant, dans son principe, la mise en place du régime dérogatoire de sortie d'indivision. Quant au caractère proportionné à l'objectif poursuivi des mesures proposées, elle a estimé que l'Assemblée nationale, en imposant une notification du projet de vente ou de partage par acte extrajudiciaire à tous les indivisaires, en renforçant les modalités de publicité du projet et en renversant la charge de la saisine du juge en cas d'opposition d'un indivisaire minoritaire au projet, avait apporté de solides garanties, qui s'ajoutaient au caractère temporaire du dispositif créé. Aussi la commission des lois a-t-elle entendu s'inscrire dans la continuité des travaux engagés, en proposant des modifications de nature à renforcer encore l'efficacité du dispositif tout en lui apportant de nouvelles garanties en termes de sécurité juridique. elle a étendu l'application du dispositif dérogatoire de sortie d'indivision aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Elle a ensuite prévu qu'il s'appliquerait seulement aux successions ouvertes depuis plus de dix ans, au lieu de cinq ans, pour permettre aux héritiers d'exercer pleinement les actions

ou l'option successorale qui peut être exercée par l'héritier dans ce même délai. Enfin, par souci de cohérence, la commission a modifié la majorité requise pour effectuer des actes d'administration ou de gestion, jusqu'à présent fixée à deux tiers des droits indivis, pour éviter qu'il ne soit plus difficile d'effectuer ces actes que de procéder à des actes de disposition. Je rappelle que la proposition de loi autorise la vente ou le partage du bien sur l'initiative des indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis seulement. À l'article 2, en cas de projet de vente du bien à une personne étrangère à l'indivision, la commission a prévu la possibilité, pour tout indivisaire qui le souhaiterait, d'exercer un droit de préemption pour se porter acquéreur du bien aux prix et conditions de la cession projetée. Pour encourager les héritiers à partager les biens indivis, elle a introduit dans le texte un nouvel article 2 , tendant à mettre en place une exonération du droit de partage de 2,5 % pour les immeubles situés dans les territoires ultramarins concernés par le dispositif dérogatoire de sortie d'indivision. Sur l'initiative de notre collègue Lana Tetuanui, elle a également introduit dans le texte un nouvel article 5 qui consacre la possibilité de procéder, en Polynésie française, à un partage du bien par souche, quand le partage par tête est rendu impossible en raison, notamment, du nombre d'héritiers ou de l'ancienneté de la succession. À l'article 5, la commission a étendu, aux autres collectivités ultramarines concernées par le texte, l'application du mécanisme créé au bénéfice de la Polynésie française, consistant à permettre au conjoint survivant ou à un héritier copropriétaire de bénéficier de l'attribution préférentielle du bien sur lequel il a établi sa résidence. La commission a procédé à la même extension à l'article 6, à l'article 6, s'agissant du dispositif visant à empêcher la remise en cause d'un partage judiciaire transcrit ou exécuté par un héritier omis à la suite d'une erreur ou d'une ignorance. Bien consciente que ce texte ne résoudra pas, à lui seul, les difficultés foncières des territoires ultramarins, la commission a néanmoins estimé qu'il pourrait constituer un outil intéressant de sécurisation du foncier s'il était associé à d'autres initiatives, comme

Madame la présidente, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, les auteurs de la proposition de loi, tout comme les membres de la commission des lois, ont eu raison de rester prudents

outre-mer. Il faut non seulement respecter des identités et des rapports particuliers à la terre, mais aussi concilier cette mobilisation du foncier, sans laquelle aucun développement n'est possible, avec une organisation sociale dans laquelle la famille et la mise en valeur de biens communs ont une tout autre place et une et une tout autre forme qu'en métropole. Comme le rappelle, dans son rapport d'information de juin 2016, la délégation sénatoriale à l'outre-mer : « [ ...] par-delà les différences, l'attachement à la terre, la terre des ancêtres, constitue un trait commun à l'ensemble des outre-mer. Il s'agit d'un lien viscéral à forte charge symbolique et affective. La terre, pivot de l'organisation économique et sociale des sociétés ultramarines, voit son mode de gouvernance dominé par les principes de la solidarité et du consensus. d'ailleurs pas si étranger à nos réalités métropolitaines ! C'est le type de problèmes que l'on peut rencontrer lorsque l'on entend réformer la législation relative aux biens sectionaux communaux. ! Dans certains départements, ces derniers constituent toujours une forme d'exploitation collective bien vivante, alors que dans d'autres, ils ne sont qu'une survivance paralysante-

Ne pensant pas utile de répéter ce qui vient d'être excellemment exposé par Mme la garde des sceaux et par notre rapporteur, je me contenterai d'approuver les propositions qui nous sont faites,

et l'exonération temporaire du droit de partage des opérations prévues par le dispositif dérogatoire. J'ai cru comprendre que le Gouvernement était opposé à cette

Madame la présidente, madame la garde des sceaux, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, si le sujet qui nous occupe aujourd'hui paraît, au premier abord, étroitement technique, il n'en est pas moins essentiel, en ce qu'il touche directement au quotidien de nos concitoyens d'outre-mer. Le foncier et l'indivision constituent deux problématiques majeures auxquelles sont confrontées les collectivités d'outre-mer et, à travers elles, leurs populations. Plus que de mesures juridico-financières, il est ici question de mesures sociales, avec des familles qui, ne pouvant se loger, se retrouvent bloquées dans leurs projets de vie. En Martinique, par exemple, 40 % du parc immobilier est en indivision. Ce seuil ne nous inquiéterait pas outre mesure si la conception traditionnellement communautaire de la propriété et la forte émigration des indivisaires vers la métropole n'avaient pas conduit au blocage de la situation de nombreux biens. Ces derniers étant parfois absents ou réticents à la cession, les indivisions « bloquées » se sont en effet multipliées. Prenez le village mahorais de Chiconi, où deux indivisions de 75 et 81 hectares représentent à elles seules les trois quarts de la surface immobilière locative locale. C'est énorme Qui plus est lorsque l'une d'elles regroupe 69 indivisaires. Plus préoccupant encore, certaines indivisions en Polynésie française sont à présent centenaires et concernent parfois jusqu'à un millier de personnes, sans que l'on puisse, en l'état actuel du droit, traiter ces dossiers de façon satisfaisante. Certes, les tribunaux locaux ont su s'adapter, dégageant en quelque sorte leur propre droit, et appliquant des principes variés comme la souche familiale, le droit au retour ou encore l'attribution préférentielle. Je vous passerai enfin l'énumération des conséquences négatives qu'entraîne ce phénomène d'indivision et que les auteurs de la présente proposition de loi ont parfaitement identifiées. Je vous dirai simplement qu'il est aujourd'hui urgent que nous libérions le foncier en outre-mer. Cette libération doit être durable, stable et, surtout, assise sur de solides bases légales. En tant que représentants des collectivités locales et des territoires, nous devons être vigilants à la situation de l'outre-mer. C'est ce à quoi s'attache le texte de nos homologues du groupe Nouvelle Gauche à l'Assemblée nationale, et c'est ce à quoi a veillé la commission des lois du Sénat. Je salue d'ailleurs le travail de la commission, qui a su, avec acuité, amender le texte afin de le rendre plus équilibré et plus efficient. En effet, ce n'est pas chose aisée que de parvenir à un texte qui n'empiète pas de façon disproportionnée sur les droits de propriété des indivisaires minoritaires, tout en renforçant l'efficacité du dispositif juridique. Bien considérée, cette proposition de loi permet une stabilisation des droits de propriété de la majorité des indivisaires, sans rendre pour autant impuissants ceux qui seraient hostiles à la vente. Il s'agit d'un bel équilibre trouvé. Aussi vais-je revenir sur ce qui a été décidé en commission. Le champ d'application des articles 1, 5 et 6 a été opportunément étendu par la commission afin de couvrir des collectivités ultramarines jusqu'ici oubliées par la proposition de loi. Il s'agit d'une bonne chose, car, si la situation n'est pas identique d'une île à l'autre, la libération du foncier doit se faire pour l'ensemble de l'outre-mer. L'article 1 prévoit un dispositif dérogatoire de sortie d'indivision aux successions ouvertes depuis plus de dix ans- et non plus cinq ans, comme le prévoyait le texte transmis par l'Assemblée. Ce nouveau délai devrait opportunément permettre de rendre le dispositif compatible avec certaines actions ouvertes par le code civil s'inscrivant dans des délais plus longs. Tel est ainsi le cas de l'action en possession d'état pour établir une filiation filiation avec le, qui se prescrit par dix ans, ou encore de l'option successorale, qui peut être exercée par l'héritier dans ce même délai. La proposition de loi autorise par ailleurs la vente ou le partage du bien sur l'initiative des indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis seulement, ce qui n'était pas cohérent avec l'exigence, à présent supprimée, d'une majorité fixée à deux tiers. Ces deux modifications apportées en commission montrent le sérieux et la pertinence du travail sénatorial. Plus fondamentalement, nous approuvons les dispositions spécifiques prévues à l'article 1, afin d'empêcher qu'une vente ne s'opère lorsqu'elle risquerait de léser certaines personnes vulnérables. Cette mesure procède du bon sens. En prévoyant expressément, à l'article 2, la possibilité pour tout indivisaire qui le souhaiterait d'exercer un droit de préemption pour se porter acquéreur du bien, aux prix et conditions de la cession projetée, la commission a par ailleurs su prendre en compte l'histoire de terres qui, pour les familles concernées, font l'objet d'un attachement charnel, au plus grand bénéfice de la culture locale. Et parce qu'il était nécessaire de mettre fin au rôle bloquant des indivisaires minoritaires, c'est une bonne chose que la commission des lois ait supprimé la notion de « présomption de consentement », estimant qu'il était plus pertinent de prévoir que la vente ou le partage du bien leur serait « opposable Ainsi, un indivisaire seul qui refuse de prêter son concours à la vente ou au partage sans pour autant s'y opposer ne bloquera plus l'ensemble du processus et sera présumé consentir à la vente. De même, l'ajout de l'article 2 est bienvenu dans l'optique de libération du foncier que j'évoquais. Je profite du temps qui m'est donné pour saluer notre collègue Lana Tetuanui, dont le travail a conduit à l'introduction de l'article 5 A, même si le sujet, je l'avoue, reste très complexe. Il serait désormais possible, en Polynésie, de procéder à un partage du bien par souche, quand le partage par tête est rendu impossible en raison notamment du nombre d'héritiers ou de l'ancienneté de la succession. Cet article fait ainsi écho aux attentes de la cour d'appel de Papeete et se conforme utilement au code de procédure civile de la Polynésie française. Ce texte serait en définitive une avancée importante. Il devrait permettre aux collectivités de conduire une politique du logement plus efficace et plus juste.

nous voilà réunis pour examiner une proposition de loi présentée il y a quelques semaines à l'Assemblée nationale. Nous voilà réunis pour donner du sens, de la suite, du corps à une volonté longtemps exprimée par plus d'un avant moi, et notamment Aimé Césaire, député de la Martinique, d'une exigence légitime de différenciation. D'ailleurs, c'est avec un certain bonheur que je constate que ce mot- heureux -est désormais adopté par le Président de la République et son gouvernement à l'endroit de nos pays. déplaise aux adeptes de l'uniformité de la République, ladite outre-mer est différente ! Différente par son histoire, différente par ses peuplements, différente par les affres et les traces laissées par ses migrations souvent imposées, différente par sa- que dis-je ! -, par ses cultures, ses moeurs, marquée par un vécu ô combien douloureux écrit à l'encre indélébile, une encre aux couleurs d'inégalités rapiécées, d'injustices banalisées, d'oppressions sanglantes. Pas simple, cette histoire. Pas simple du tout ! Et c'est parce qu'elle n'est pas simple que nous sommes là aujourd'hui. C'est parce qu'elle n'est pas simple que l'histoire- son histoire -nous convoque aujourd'hui ici, solennellement, pour exprimer ensemble cette évidence : celle de la différence. Le pouvoir hélas ! a souvent nié cette différence et a maintes et maintes fois souhaité que, y compris par la force sanglante, ces pays se couchent, se plient dans le moule qui muselle toute initiative, toute conquête, toute émancipation. Le cheminement pour le progrès humain a été long, très long, y compris après que, l'esclavage une fois aboli, a enfin commencé une quête de la reconnaissance d'une humanité. Oui, d'une humanité Et c'est dans cette humanité jeune finalement, vieille de quelques décennies, d'il y a à peine un siècle et demi, que l'homme de ladite outre-mer tente durement, laborieusement, de trouver sa place, d'exister, enfin de survivre pour exister. La notion de propriété est une histoire vieille pour la vieille Europe conquérante, mais tellement récente pour nous. Lâché dans un nouveau monde déshumanisé, il restera à l'ancien esclave à tout faire, tout construire. Être propriétaire ? Souvent une chimère. Avec quoi ? Sans instruction, sans moyens, rémunéré dès lors certes, mais à quel prix : trois francs six sous Alors, quand le fruit du labeur le permet enfin, sou par sou, goutte de sueur par goutte de sueur, le bien acquis, la petite case, les trois acres de terre cultivable deviennent tellement chers, tellement précieux, tellement pleins de valeur qu'il n'est pas envisageable de régler une quelconque succession avant le jour du départ pour l'au-delà. Ce qui est rare est cher, ce qui est rare a du prix Pour rajouter à cette complexité de la différence, cent ans après l'abolition de l'esclavage, le pouvoir organise la migration, une nouvelle, une de plus. Il faut « dégonfler » au plus vite ces îles hideuses, pauvres et misérables, qui commencent à gronder. Vingt années de migration forcée vers ladite métropole censée être le nouvel eldorado voient arriver ces oubliés de l'histoire par dizaines de milliers : les convoqués du BUMIDOM, les enfants de la Creuse sont les exilés d'un nouveau genre. On avait choisi le plus facile, le plus ignoble aussi. On avait choisi d'ignorer cette humanité, de ne pas l'affronter avec courage et réalité. On dépossède encore une fois. Une fois de plus, une fois de trop Les enfants partent par milliers, par dizaines de milliers, encouragés y compris par leurs parents qui rêvent pour eux d'un avenir meilleur. Beaucoup ne reviennent pas, fuient ces pays dans lesquels les souvenirs ont souvent la couleur de leur peau. Explosées partout dans le monde, nombreuses, très nombreuses en France, les générations se succèdent sans se raccrocher pour autant à un pays dont beaucoup ignorent tout. Et les biens sont restés là, en l'état. Plus personne pour s'en occuper. L'écheveau emmêlé de la succession devient une affaire inextricable. Les héritiers en cascade ont du mal à être repérés, à être identifiés. Les familles s'affrontent, des drames surviennent, et la solution est souvent l'abandon. On abandonne pour laisser à l'univers public son lot de désolation : squats, réserves naturelles nombreuses pour le moustique tigre, qui sème dengue, chikungunya. Les villes sont défigurées par ces masures, ces terrains en friche. Pour le pays que je connais le mieux, la Martinique, dans certaines communes on peut compter jusqu'à un taux de 83 % de cas d'indivisions non réglées,

Le contexte que je me suis appliquée à décrire dans mon exposé en est la cause réelle et sérieuse. Alors, comment faire pour accompagner un règlement plus rapide de ces situations, qui posent de véritables problèmes à la santé publique, à la préservation sanitaire, mais aussi à l'ordre et à la cohésion familiale ? Oui, comment faire, sinon faire différent ? Comment faire, sinon coller à un contexte singulier et particulier ? J'en profite pour remercier le Gouvernement, et particulièrement Annick Girardin, qui a pu se rendre compte de la situation sur le terrain, mais aussi votre ministère, madame la garde des sceaux, qui a compris que le droit commun ne pouvait correspondre à cette réalité. Il faudra donc déroger. L'initiateur de cette proposition de loi, le député Serge Letchimy, a proposé que cela se fasse sur dix ans, le temps nécessaire pour un sérieux coup de plumeau. Nous lui devons notre confiance. Il sait de quoi il parle, il maîtrise cette matière. Docteur en urbanisme, le député Letchimy possède à son actif des dizaines de procédures de réhabilitation de quartiers entiers. Son histoire a d'ailleurs été retracée sous la plume d'un brillant écrivain martiniquais, Patrick Chamoiseau, dans un ouvrage qui a obtenu le prestigieux prix littéraire Goncourt. Maire de Fort-de-France pendant dix ans, Serge Letchimy avait fait de ces biens abandonnés une véritable croisade. Pour l'avoir accompagné dans ses mandatures municipales en tant qu'adjointe en charge de la sécurité, j'ai eu pour un seul quartier- je dis bien un seul -, sur les cent trente que compte Fort-de-France, à traiter le cas de pas moins de 300 maisons qui relèvent de cette situation de succession non réglée. Alors, c'est en toute connaissance de cause et pour ne pas rester, pour citer Césaire, « les bras croisés dans l'attitude stérile du spectateur », qu'il a pris l'initiative de proposer cette heureuse dérogation. Il n'est pas du genre à capituler devant la difficulté, devant le cadre qui étrangle, qui enserre. Il faut en permanence inventer. Il a été pour cela aidé dans sa tâche par des professionnels des questions de propriété, notaires, établis ou en devenir. J'ai à cette occasion une pensée particulière pour l'une d'entre eux, Samantha Chevrolat, à laquelle je rends un hommage appuyé aujourd'hui pour son engagement. Cette loi est attendue. Nos populations piaffent d'impatience. Le parquet de Fort-de-France a même salué l'initiative lors de sa rentrée solennelle pour dire et souligner la fluidité qu'elle provoquera dans de nombreuses procédures, en particulier dans nos tribunaux engorgés. Des réunions se tiennent déjà partout. Ce n'est

Au moment où je vous parle, aujourd'hui 4 avril, ce dernier est reçu, car réclamé, en Guadeloupe, au Gosier, pour une réunion publique au côté de deux autres députés, Max Mathiasin et Justine Benin, pour dire et redire l'urgence de cette disposition. Alors, aujourd'hui, on parlera beaucoup de droit, je le sais, on fera référence à l'article le meilleur, le plus rigide aussi parfois. On ira chercher certainement le détail là où se cache le diable pour encadrer, « enrichir » comme on dit. Le débat doit avoir lieu, il est légitime et normal et j'y tiens, avec le plus grand respect pour l'expression de toutes les opinions. Les amendements suscités sont certes légitimes et nourrissent en quelque sorte l'idée que cette loi était finalement espérée. Mais ne perdons pas de vue, en sagesse, l'essentiel. Moi, j'ai eu envie de vous parler de la réalité d'une élue de ladite République d'outre-mer, celle dont les ancêtres ont dû souvent « marronner », autrement dit faire autrement, faire différent, pour faire entendre leur cause. Oui, au fond de moi, j'ai la force et la conviction que le droit sans la reconnaissance d'une humanité réelle et assumée peut mal, peut injuste, peut maladroit. Colbert, qui me surplombe ici en ce moment, avait lui aussi choisi le droit en son temps, le droit bien écrit, le droit face à l'humanité, l'humanité différente, au travers du Code noir. En assurant à des milliers de familles décomposées, recomposées, triturées, tout en garantissant la stricte préservation de leurs droits, une fluidité contextuelle, conjoncturelle au règlement de leurs déboires, la République aura signifié son entrée magistrale dans cette revendication de la différenciation. Les meilleures lois pour l'outre-mer seront désormais celles qui préserveront ce droit à la reconnaissance d'une singularité que nous ne demandons qu'à assumer. Aux collectivités régies par l'article 74 de la Constitution qui ont choisi de s'inscrire dans la dynamique de cette proposition de loi, je ne peux que dire : bienvenue ! Nos histoires communes ne sauraient être étranglées par le fétichisme d'un article de la Constitution. Assemblons donc tout ce qui se ressemble. Mais ne perdons jamais de vue que nous traitons là de questions urgentes, qui faciliteront le quotidien aussi bien des maires, des élus, des responsables de l'État que de milliers, de dizaines de milliers de familles en attente dans les couloirs encombrés des tribunaux- souvent sous-dotés en moyens -de la République. Cette résolution n'est pas destinée à devenir le point de règlement de tous les sujets liés à l'indivision. Il s'agit d'un sujet particulier. Un petit proverbe de chez nous nous rappelle nous nous rappelle :- autrement dit : l'excès en tout nuit. Ne noyons pas l'essence de ce texte, considérons-le comme une boîte à outils pertinente. La demande est simple simple : de quoi s'agit-il en fait ? Permettre aux indivisaires de passer de l'unanimité requise pour un partage à la majorité ; permettre aux successions ouvertes depuis plus de cinq ans de procéder à la vente ou au partage du bien ; permettre aux notaires, sans passer par les tribunaux, tellement engorgés, d'accomplir les actes en prenant toutes les précautions formelles

les situations d'indivision sont devenues inextricables. Cet état de fait contribue au gel du foncier disponible sur des territoires insulaires où celui-ci est rare. L'activité économique y est ainsi entravée. Cette indivision durable et généralisée trouve son origine dans des raisons propres à chaque territoire, notamment le recours peu fréquent ou tardif aux notaires, la méfiance des familles et la crainte de spoliation, le coût des mutations et taxes sur les successions pour des familles souvent modestes. Dès lors, dans les territoires ultramarins, il est fréquent de constater des successions non réglées sur plusieurs générations et des partages non faits ou non enregistrés selon les règles, entre plusieurs dizaines et parfois plusieurs centaines d'ayants droit indivisaires Ainsi, à Mayotte, que connaît bien notre rapporteur, le territoire de certaines communes se trouve presque intégralement en situation d'indivision. En Polynésie française, les nombreuses indivisions réunissent parfois des centaines d'indivisaires à la faveur de successions non liquidées depuis quatre ou cinq générations. En Martinique, 26 % du foncier est géré en indivision et 14 % supplémentaires correspondent à des successions ouvertes. Face à cette situation particulière du foncier ultramarin, très bien décrite dans le rapport d'information de la délégation sénatoriale à l'outre-mer, le législateur a souhaité intervenir pour adapter les règles du droit commun aux caractéristiques et contraintes spécifiques de ces territoires d'outre-mer en mettant en place un dispositif dérogatoire et temporaire de sortie d'indivision applicable jusqu'au 31 décembre 2028. La commission des lois du Sénat, qui s'est inscrite dans la continuité des travaux engagés par l'Assemblée nationale, a souhaité renforcer bien plus encore l'équilibre entre efficacité et sécurité juridique du dispositif. Je m'en réjouis. À l'article 1, la commission des lois a étendu l'application du dispositif dérogatoire aux collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Elle a ensuite prévu qu'il ne s'appliquerait qu'aux successions ouvertes depuis plus de dix ans et non pas aux successions ouvertes depuis plus de cinq ans, pour permettre aux héritiers d'exercer pleinement les actions qui leur sont ouvertes par le code civil. Enfin, elle a mis en cohérence la majorité requise pour effectuer les actes d'administration et de gestion sur un bien détenu en indivision avec la nouvelle majorité retenue par le présent texte pour vendre ou partager le bien plus de la moitié des droits indivis. À l'article 2, en cas de projet de vente du bien à une personne étrangère à l'indivision, la commission des lois a prévu la possibilité pour tout indivisaire qui le souhaiterait d'exercer un droit de préemption pour se porter acquéreur du bien aux prix et conditions de la cession projetée. Elle a ensuite supprimé la notion de présomption de consentement au projet de l'indivisaire qui ne se serait pas manifesté, estimant qu'il était plus pertinent de prévoir que la vente ou le partage du bien lui serait opposable. Par ailleurs, la commission, afin d'encourager les héritiers à partager les biens indivis, a introduit un nouvel article 2 qui met en place une exonération de droit de partage de 2,5 % pour les immeubles situés dans les territoires ultramarins concernés par le dispositif dérogatoire de sortie d'indivision.

en Polynésie française, à un partage du bien par souche, quand le partage par tête est rendu impossible en raison, notamment, du nombre d'héritiers ou de l'ancienneté de la succession. À l'article 5, la commission a étendu, aux autres collectivités ultramarines concernées par le texte, l'application du mécanisme créé au bénéfice de la Polynésie française, consistant à permettre au conjoint survivant ou à un héritier copropriétaire de bénéficier de l'attribution préférentielle du bien, en démontrant qu'il y a sa résidence de manière continue, paisible et publique depuis plus de dix ans au moment de l'introduction de la demande de partage en justice. Enfin, la commission des lois a procédé à la même extension, à l'article 6, s'agissant du dispositif visant à empêcher la remise en cause d'un partage judiciaire transcrit ou exécuté par un héritier omis à la suite d'une erreur ou d'une ignorance, en limitant son action à la faculté de demander de recevoir sa part, soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage. Avant de conclure, je souhaite saluer, à cette tribune, le travail effectué par notre rapporteur sur un sujet d'une grande complexité. Madame la ministre, mes chers collègues, conscient que cette proposition de loi ainsi enrichie par la commission des lois du Sénat ne résoudra pas, à elle seule, les importantes difficultés foncières des territoires ultramarins, notre groupe estime toutefois qu'elle constitue un outil très utile de sécurisation du foncier.

Madame la présidente, madame la garde des sceaux, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, cette proposition de loi peut susciter d'emblée trois interrogations de la part de nos concitoyens ou même de nos collègues quelle est la nécessité de légiférer spécifiquement sur la problématique de l'indivision ? pourquoi uniquement en outre-mer ? et pour quels résultats ? Les réponses, mes chers collègues, figurent dans le rapport de mission de notre délégation à l'outre-mer. En effet, cette proposition de loi s'inspire très largement du rapport d'information

Sous le titre « Une caractéristique de la situation foncière des outre-mer », M. le rapporteur nous livrait cette phrase tout à fait éclairante Le manque de sécurité de la propriété privée se manifeste dans la conjonction d'une carence de titrement et d'une indivision endémique. » Tous les territoires ultramarins connaissent en effet ces problématiques, avec des degrés variables de complexité. Tout d'abord, la carence de titrement : de nombreux biens immobiliers ou terrains sont détenus sans titre de propriété ou sans document juridique. Il est donc extrêmement difficile aujourd'hui de « régulariser » ces situations, dès lors qu'un droit de propriété est contesté. À cela s'ajoute une autre difficulté, qui se cumule souvent à la première : l'indivision, qui est largement répandue en outre-mer. Ainsi, nombreux sont les terrains et les biens qui appartiennent non pas à une personne seule, mais à une famille. Pour réaliser une transaction immobilière, il faut donc l'accord de l'ensemble des membres de la famille, ce qui peut aisément représenter plus de dix personnes.

quel est l'apport de la proposition de loi de notre collègue député Serge Letchimy ? Le texte initial a connu des améliorations tant à l'Assemblée nationale qu'au sein de notre commission des lois. Pour citer les notaires de Saint-Martin que j'ai pris le soin de consulter en amont, « il était juridiquement surprenant qu'un texte dérogatoire fixe une majorité à 51 % pour les actes pour les actes de disposition les plus graves- partages et ventes -et une majorité de deux tiers pour les actes d'administration ». Je me félicite donc de l'harmonisation à 51 % dans les deux cas ou encore de l'attribution préférentielle introduite par l'article 5. Cependant cette proposition de loi présente des limites, car il est extrêmement fréquent que les indivisaires soient très nombreux et que plusieurs d'entre eux aient quitté le territoire et que les familles soient éclatées de par le monde. Or il y a parfois méconnaissance de l'identité et de la localisation précises de certains indivisaires. Aussi, afin de donner plus de chances aux indivisaires d'exprimer leur désaccord éventuel,

Un autre problème qui n'a pas du tout été abordé est celui des indivisaires en pleine capacité juridique, mais « incapables » dans la réalité. Je pense aux personnes en rupture familiale, aux personnes sous influence de substances addictives, mais aussi aux personnes en situation de handicap. Je sais que la situation des majeurs incapables est prévue par la loi, notamment par le placement sous tutelle ou sous curatelle. Mais, à Saint-Martin, les familles n'ont pas culturellement pris l'habitude de systématiquement signaler leurs proches incapables ou ne font pas les démarches administratives nécessaires. Ce n'est que par un long processus d'acceptation psychologique et culturelle que ce sujet évoluera dans les territoires ultramarins, mais en attendant, il serait pourtant nécessaire de prendre des mesures dérogatoires et protectrices. Il est indiscutable, mes chers collègues, que cette proposition de loi représente une avancée utile et nécessaire pour nos territoires ultramarins. C'est la raison pour laquelle je suis favorable à son application à Saint-Martin, ce qui n'était prévu ni dans la version initiale ni dans le texte issu des travaux de l'Assemblée nationale. Cependant, loi ouvre également la voie à d'autres difficultés comme le règlement financier des droits de succession pour des familles souvent largement précarisées. Car il s'agit généralement non pas de régler une succession directe, mais de traiter une suite de successions non réglées. Nous pensions également à tort que l'indivision permettait de protéger le patrimoine familial, mais il ne faudrait pas non plus qu'il ouvre trop facilement la porte à la spéculation immobilière et foncière.

Les pratiques traditionnelles et familiales en outre-mer sont la raison d'une indivision bien plus importante qu'en métropole. Cette spécificité territoriale, conjuguée à une insuffisance des registres et des actes notariés, multiplie les situations de blocage des successions de biens. La forte émigration des indivisaires n'arrange pas les choses, puisque ceux-ci sont parfois inconnus, absents ou réticents à la cession du bien. Par conséquent, les successions prennent de nombreuses années et donnent lieu à des situations aberrantes, avec des dossiers parfois centenaires à la suite d'une cascade de successions. S'ajoutent au grave problème d'indisponibilité du foncier des conséquences sur le plan sanitaire : les bâtiments non entretenus deviennent de véritables nids à épidémie où prolifèrent les moustiques vecteurs de la dengue, de la fièvre jaune et du chikungunya. Il faut aussi relever les répercussions en termes d'aménagement ainsi que de rentrées fiscales pour les collectivités, ce qui a pour effet de compromettre le développement économique. Les tribunaux locaux ont développé une jurisprudence au fil des situations rencontrées de manière à réduire autant que possible le nombre de litiges. Pour autant, et malgré tous leurs efforts, ce n'est pas suffisant face à l'ampleur du problème. Il fallait remédier à cette situation. C'est pourquoi la présente proposition de loi est la bienvenue. L'article 1 dispose que les indivisaires titulaires de plus de la moitié en pleine propriété des droits indivis pourront désormais vendre, alors qu'il fallait jusqu'à présent obtenir l'accord de toutes les personnes Imaginez la situation lorsque cela concerne une famille nombreuse, avec une succession qui s'éternise. Une sécurité juridique a été prévue : il faudra attendre cinq années après la succession pour faire valoir ce droit et le notaire interviendra systématiquement, ce qui n'était pas toujours le cas auparavant. Nul ne pourra arbitrairement, au lendemain de l'ouverture de la succession, décider de bloquer la situation et prendre au dépourvu les autres indivisaires sans laisser le temps de trouver un compromis. De plus, ce nouveau régime serait valable pour une période de dix ans, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2028, de manière à ouvrir provisoirement ces possibilités et à permettre par dérogation le déblocage de nombreuses situations. Il s'agit en quelque sorte d'étendre et d'adapter aux territoires d'outre-mer la « solution corse » de la loi du 6 mars 2017. Les nouvelles dispositions, en outre, ne laissent pas impuissant l'indivisaire hostile à la vente ou au partage, puisque celui-ci pourra faire connaître son hostilité sous trois mois. Il reviendra alors au tribunal de grande instance de trancher après saisine des indivisaires majoritaires. Des dispositions Des dispositions spécifiques ont également été comprises dans cet article afin d'empêcher qu'une vente s'opère lorsqu'elle risquerait de léser certaines personnes vulnérables. Cela concerne les locaux d'habitation occupés par des conjoints survivants au défunt, des indivisaires mineurs et majeurs protégés ou des indivisaires présumés absents. De telles mesures,, peuvent paraître constituer un empiètement sur les droits de propriété des indivisaires mis en minorité lors de la prise de décision. Mais elles sont au contraire un moyen de stabiliser la situation des droits de propriété de la majorité des indivisaires. Une telle mesure garantit aussi la paix publique, parce qu'elle apaise les familles, qui peuvent parfois malheureusement se déchirer à la suite d'une succession. C'est pourquoi je voterai en faveur de la proposition de loi visant à faciliter la sortie de l'indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer, qui me semble utile pour répondre à la situation. La parole

En Marche. Madame la présidente, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, nous sommes aujourd'hui appelés à légiférer sur une proposition de loi visant à apporter une solution à un problème très ancien dans nos régions l'indivision successorale. Pourquoi viser précisément les territoires ultramarins ? Parce que, dans ces collectivités, l'accès à la propriété, fort difficile, est encore aggravé par ce système d'indivision.

dans la mesure où tous les héritiers doivent être rassemblés pour qu'une décision soit prise au sujet d'un bien immobilier hérité- la vente, par exemple -, le bien reste souvent inutilisé, à l'abandon, et les ressources qu'auraient pu en tirer les héritiers restent lettre morte. Cette situation est due à un état du droit archaïque qui a besoin d'une simplification. C'est cette simplification que tend à apporter la présente proposition de loi. M. le député de la Martinique Serge Letchimy, auteur de la proposition de loi, a, par exemple, souligné qu'en Guadeloupe les familles, connaissant mal leurs droits en la matière, recourent peu au notaire pour la transmission et ignorent les règles régissant l'indivision. Ce processus est accentué par un manque de confiance des citoyens ultramarins dans le droit français. On est donc face à une véritable paralysie foncière. En Martinique, par exemple, plus de 40 % du foncier est gelé pour cause d'indivision successorale. Les conséquences ne sont pas seulement néfastes pour le foncier. L'indivision successorale signifie aussi un engorgement des juridictions d'outre-mer dû au contentieux successoral. Aussi, le texte examiné aujourd'hui, adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, devrait rencontrer la même approbation au Sénat, puisque, d'une part, il tend à autoriser les indivisaires représentant la majorité des droits indivis à provoquer la vente ou le partage et, d'autre part, préciser qu'un indivisaire opposé au projet d'acte notifié saisit le tribunal de grande instance à fin de partage judiciaire dans les conditions de droit commun. En somme, il s'agit d'un nouvel outil destiné à résoudre une grande partie des difficultés foncières. Si l'on devait le résumer en une phrase, je dirais que tout repose sur la dérogation à la règle de l'unanimité en matière de consentement. Il s'agit en effet d'adapter la procédure aux spécificités des territoires ultramarins. Alors que, dans l'Hexagone, il est souvent aisé de réunir les indivisaires lors du partage des biens hérités, il en va tout autrement en outre-mer, où les familles sont par ailleurs très nombreuses. Dans ces situations, l'article 73 de la Constitution autorise le législateur à intervenir pour adapter les règles de droit commun aux caractéristiques et aux contraintes particulières de ces territoires, habituellement soumis à la règle de l'identité législative. En premier lieu, je souhaiterais souligner que le dispositif dérogatoire prévu par la présente proposition de loi est temporaire. L'article 1 vise en effet à prévoir que les dispositions du texte seront valables jusqu'au 31 décembre 2028. Il s'agit, en fait, d'apporter une réponse rapide à une situation gangrenée depuis des années. Dans la décennie qui vient, nous allons pouvoir réfléchir à une solution pérenne pour le foncier en outre-mer. Autre point important : le droit de propriété n'est pas remis en cause par le présent texte. Ce droit, garanti par les articles 2 et 17 de la Constitution, ne peut être limité, sauf s'il s'agit d'un motif d'intérêt général. Or la dérogation au droit commun prévue par la proposition de loi se justifie par un motif d'intérêt général et par le caractère proportionné à l'objectif visé par les mesures proposées, notamment en imposant une notification du projet de vente ou de partage par acte extrajudiciaire à tous les indivisaires, en renforçant les modalités de publicité du projet et en renversant la charge de la saisine du juge en cas d'opposition d'un indivisaire minoritaire au projet. En second lieu, je voudrais saluer le travail de la commission des lois du Sénat, qui, tout en restant fidèle à l'esprit du texte, l'a rendu plus efficace. Ainsi, à l'article 1, elle a étendu l'application du dispositif dérogatoire de sortie d'indivision à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Elle a ensuite décidé que ce dispositif ne s'appliquerait qu'aux successions ouvertes depuis plus de dix ans- et non cinq ans comme c'était le cas dans le texte initial -afin de permettre aux héritiers d'exercer pleinement les actions qui sont prévues par le code civil. Enfin, le texte examiné aujourd'hui, tel que modifié par la commission, prévoit que la majorité requise pour effectuer des actes d'administration ou de gestion n'est pas des deux tiers, mais est simplement de la moitié. Autre mesure importante : à l'article 5, la commission a étendu aux autres collectivités ultramarines concernées par le texte l'application du mécanisme créé au bénéfice de la Polynésie française. Ainsi, le conjoint survivant ou l'héritier copropriétaire peut désormais bénéficier de l'attribution préférentielle du bien sur lequel il a établi sa résidence. De même, à l'article 6, le dispositif visant à empêcher la remise en cause d'un partage judiciaire transcrit ou exécuté a été étendu à toutes les collectivités. Le présent texte constitue donc une avancée majeure dans la résolution du problème foncier en outre-mer. Charge au législateur de poursuivre le travail amorcé : le rapport de M. le vice-président du Sénat et sénateur de Mayotte, Thani Mohamed Soilihi, est d'ailleurs éclairant. Il propose, par exemple, la mise en place de groupements d'intérêt public ayant pour objet la reconstitution des titres de propriété. Pour toutes ces raisons, nous voterons ce texte de loi, car, comme l'a relevé Mme la ministre des outre-mer, Annick Girardin, il constitue un « premier aboutissement des travaux menés avec le Gouvernement pour porter une ambition commune ultramarine

En droit civil, l'indivision permet le maintien pour une certaine durée de l'unité d'un bien ou d'un ensemble de biens après la mort de son propriétaire : le bien est donc « indivis ». Élu de Loire-Atlantique, je peux témoigner de la complexité de l'indivision, qui répond à une situation unique en France. Par les lettres patentes accordées par le roi Louis XVI, le 28 janvier 1784, les riverains du marais de Brière- 7 000 hectares -se voient reconnaître la « propriété, possession et jouissance commune et publique » de la Grande Brière Mottière, c'est-à-dire une propriété originale puisqu'elle est collective, indivise et inaliénable. Aujourd'hui encore, les Briérons continuent à jouir de cette propriété et à gérer eux-mêmes leur marais. Comme nous le savons tous, les indivisaires partagent la jouissance du bien, mais ils ne peuvent décider qu'unanimement des actes de vente ou de bail commercial concernant le bien. L'héritage historique du parc immobilier ultramarin et des pratiques propres aux structures successorales et familiales de ces territoires ont conduit à une prévalence bien plus importante de l'indivision au sein du parc locatif en outre-mer qu'en métropole, allant jusqu'à 40 % en Martinique. Aussi, une conception Aussi, une conception traditionnellement communautaire de la propriété ainsi qu'une insuffisance des registres et actes notariés ont conduit au blocage de la situation de nombreux biens. Les indivisaires n'étant parfois pas tous connus, étant absents ou réticents à la cession, les indivisions « bloquées » se sont multipliées. Le résultat de ce phénomène est la multiplication de situations d'indivisions très complexes et lourdes. Il existe des biens constitués de plusieurs dizaines d'indivisaires, parfois plus de soixante et même jusqu'à mille personnes en Polynésie française. Cette situation de blocage rend difficile l'aménagement du territoire, avec notamment une complexification de la collecte de la taxe foncière, des procédures à rallonge, un engorgement des tribunaux locaux, une hausse importante du prix du foncier non indivis et un délabrement des biens indivis laissés à l'abandon. Des dispositifs permettant de sortir de l'indivision- je pense à l'article 815 du code civil -existent : prescription décennale de l'option successorale, administration par un mandataire successoral, constatation de l'état d'abandon d'une parcelle, expropriation pour cause d'intérêt public, etc. Pour autant, ces dispositions doivent être adaptées à la situation spécifique de la propriété indivise en outre-mer où les indivisaires ne sont, dans de nombreux cas, pas tous connus. En Martinique ou à Mayotte, par exemple, des mesures ponctuelles permettent de débloquer des situations inextricables. Il faut également citer les dispositions législatives suivantes : la loi du 23 juin 2006 a fait passer la majorité nécessaire aux actes d'administration aux deux tiers des indivisaires ; la loi du 13 octobre 2014 a fait passer la majorité nécessaire aux actes de disposition de terres agricoles ultramarines indivises à deux tiers des droits ; la loi du 6 mars 2017 a fait passer la majorité nécessaire aux actes de disposition des immeubles situés en Corse à deux tiers des droits. Concernant la présente proposition de loi, elle vise à débloquer la situation de nombreuses indivisions dans les territoires d'outre-mer français en permettant à la majorité absolue des indivisaires de vendre le bien. Un indivisaire absent ou solitaire déterminé à faire obstacle à une cession ne serait alors plus en mesure de paralyser durablement la situation d'un bien pour les successions ouvertes depuis au moins cinq ans. Cela pose néanmoins question sur le risque d'une atteinte au droit de propriété des indivisaires tel qu'il existe actuellement dans le cadre de la prise de décision. Mais, par ailleurs, n'a-t-on pas le devoir de stabiliser les droits de la majorité des indivisaires lorsqu'il est impossible de parvenir à un règlement amiable ? Au demeurant, la proposition de loi ne rend pas impuissant l'indivisaire hostile à la vente ; ce dernier peut faire connaître son opposition sous trois mois de la notification ou publication de la décision de vente. Les indivisaires majoritaires doivent alors saisir le tribunal de grande instance, qui autorise la vente ou le partage sous réserve que cela ne porte pas une atteinte excessive aux droits des indivisaires minoritaires. Espérons que ces différents dispositifs dérogatoires transitoires permettent de favoriser l'accès de nos compatriotes ultramarins à un logement décent et que l'accès aux terrains relance les programmes de construction de logements, pierre angulaire de l'aménagement des territoires en outre-mer comme en métropole. La gestion foncière est également de première importance pour les collectivités locales dans le cadre de l'élaboration des plans locaux d'urbanisme. L'action publique doit pouvoir s'appuyer sur des leviers efficaces pour une politique du logement efficiente. Lié à un enjeu d'intérêt public, ce texte est utile pourvu que ces solutions innovantes soient d'abord profitables aux Français d'outre-mer, attachés à leur terre, et qu'elles offrent la garantie d'une politique d'aménagement raisonnable. À l'Assemblée nationale, le groupe Les Républicains a été favorable à ce texte. Je souhaite qu'ici, au Sénat, il en soit de même. La

un accord sur les propositions formulées. M. le sénateur Collombat a salué le travail de la commission des lois. Mme la sénatrice Guidez a remarqué que le texte a été rendu plus aisé et plus efficient par ce même travail. M. le sénateur Alain Marc

et a fait un exposé extrêmement intéressant sur l'exigence légitime de la différenciation. Elle a parfaitement expliqué à quel point les principes constitutionnels bâtis dans la vieille Europe supposaient un temps d'adaptation et de compréhension

Alors que ce texte a fait consensus à l'Assemblée nationale, il se retrouve complètement dénaturé après son passage en commission des lois du Sénat. Sous couvert d'une sécurisation du dispositif, amendements ont été adoptés par la commission des lois sur ce texte. J'aurais été favorable à une sécurisation juridique du droit des propriétaires si le dispositif prévu par ce texte avait été imparfait ... Mais il me semble, eu égard aux nombreux échanges et travaux sur le sujet en amont et de sa discussion à l'Assemblée nationale, qu'il s'agit d'un texte cohérent, soucieux des droits et libertés de chacun et parfaitement équilibré. C'est d'autant plus vrai que, je tiens à le rappeler, le dispositif prévu est exceptionnel et dérogatoire, d'une durée limitée, applicable jusqu'au 31 décembre 2028, et trouve son pendant avec un intérêt public évident. Or trois dispositions adoptées en commission posent problème, notamment l'application de ce dispositif aux successions ouvertes depuis plus de dix ans. Quel sera le résultat d'une telle modification du dispositif initial ? Je rappelle quand même que ce texte avait pour vocation première de résoudre les problèmes d'aménagement posés par l'immobilisation du foncier privé. également à permettre de sécuriser les centres-bourgs et de rétablir l'ordre public en limitant, voire en éradiquant, les biens en déshérence, source d'insécurité. vocation à conforter la salubrité publique, car diminuer le nombre de bâtiments abandonnés réduirait d'autant les niches à moustiques : chikungunya, dengue et déchets sauvages. Enfin, il visait à replacer l'humain et les relations familiales dans un contexte plus apaisé quant au règlement des successions. Par conséquent, au regard des modifications apportées au texte initial et de la dénaturation complète de l'objectif initial, il est à craindre- du moins si le texte devait demeurer en l'état -que nos territoires ne subissent encore et toujours ce phénomène d'indivision sans possibilité de déblocage à court terme. La parole

au bout de sa rue ces terrains et bâtiments abandonnés, souvent squattés, finissant alors par devenir des lieux totalement délabrés mêlant nuisances et insécurité. se jouent souvent des affaires de successions dramatiques conduisant des femmes et des hommes à louer un appartement pendant que leur maison familiale tombe en ruines. J'ajoute que ce texte participe de la revitalisation des centres-bourgs, que nous appelons de tous nos voeux.

nous sommes ici tous conscients que ce texte ne résoudra pas, à lui seul, les difficultés foncières de nos territoires. Il peut néanmoins constituer un outil complémentaire pertinent pour libérer et sécuriser le foncier. Je comprends le souhait de certains de nos collègues de rendre ce dispositif aussi rapidement que possible opérationnel. Il y a urgence à agir, nous sommes tous d'accord sur ce point. Je crois néanmoins que notre rôle de législateur est aussi de voter une loi cohérente qui sécurise nos concitoyens.

toute succession ouverte depuis plus de cinq ans. La commission des lois, en portant ce délai à dix ans, a réduit fortement la portée du dispositif et a, autrement dit, affaibli cette initiative. Nous souhaitons donc en revenir au délai initial de cinq ans.

Il vise en effet à revenir au texte initial, qui prévoyait d'appliquer le dispositif dérogatoire de sortie d'indivision aux successions ouvertes depuis plus de cinq ans. La commission a préféré le rendre applicable aux successions ouvertes depuis plus de dix ans, car elle a estimé que cette durée de cinq ans n'était pas compatible avec certaines actions ouvertes aux héritiers par le code civil, comme l'action en possession d'état prévue à l'article 330 du code civil, qui permet l'établissement du lien de filiation avec le défunt dans un délai de dix ans, à l'article 780 du code civil, aux termes duquel l'héritier a dix ans pour exercer son option successorale. À cela s'ajoute la possibilité pour l'administration fiscale d'exercer un recours contre la déclaration de succession jusqu'à six ans après le décès. Dès lors, la commission a estimé peu probable que les praticiens- et je les ai auditionnés sur tous les territoires d'outre-mer conscients du risque de voir le partage ou la vente remis en cause, mettent en oeuvre le dispositif dérogatoire de sortie d'indivision avant l'expiration d'un délai de dix ans. Par ailleurs, la commission a considéré que les situations d'indivision problématiques étaient justement les plus anciennes,

du Gouvernement ? Comme l'a dit M. le rapporteur, l'amendement vise à appliquer le dispositif aux successions ouvertes depuis plus de cinq ans, délai qui était initialement prévu dans la proposition de loi et qui a été porté

quant à l'acceptation de la succession ou à la renonciation, ou encore avec le délai de droit commun des actions en matière de filiation. Toutefois, si l'objectif du texte est bien de créer un véritable choc de libération du foncier,

Je renvoie le Gouvernement à son incohérence affichée entre les deux chambres, et je demande à mon groupe et à tous ceux qui nous soutiennent de bien vouloir maintenir ce délai à cinq ans.

La commission des lois a adopté un amendement qui permet d'étendre cette majorité de 51 % aux actes de gestion et d'administration des biens indivis, qui sont actuellement soumis à la majorité des deux tiers.

Le texte que nous examinons aujourd'hui n'a pas vocation à régler tous les problèmes de succession et d'indivision. Nous avons voulu, bien au contraire, un dispositif resserré autour d'un objectif précis : faciliter les sorties d'indivision et libérer le foncier en outre-mer. Nos propositions ont été ajustées pour qu'elles puissent prospérer rapidement. Toute extension du champ du texte initial risque d'entraver son adoption définitive.

en cohérence la majorité requise pour effectuer les actes d'administration sur un bien détenu en indivision avec la nouvelle majorité retenue par le présent texte pour vendre ou partager le bien, soit plus de la moitié des droits indivis. de cette harmonisation, les auteurs de l'amendement font simplement valoir que toute extension du champ du texte initial risque d'entraver son adoption définitive. Or la commission des lois a considéré qu'il n'était pas cohérent d'exiger une majorité simple pour les actes les plus graves, alors qu'en application du droit commun les actes de gestion ou d'administration du bien nécessiteraient de recueillir l'accord des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, certes selon une procédure plus légère.

Toutefois, il pourra être observé que la réalisation d'actes d'administration, à une majorité des deux tiers, et celle de la vente, à une majorité de 51 %, ne sont pas tout à fait comparables puisque la réalisation de la vente par les indivisaires nécessite une information préalable de l'ensemble des indivisaires et une absence d'opposition expresse des indivisaires minoritaires. L'abaissement du seuil pour les actes de disposition- vente et partage -est ainsi accompagné de garanties en termes d'information et de droit d'opposition. En cas d'opposition de l'un des indivisaires minoritaires, une autorisation judiciaire préalable reste nécessaire. Par ailleurs, je rappelle que l'objet de la proposition de loi est centré sur la sortie de l'indivision et ne porte pas sur l'administration ou la gestion de l'indivision. Pour ces raisons, le Gouvernement s'en remet de nouveau à la sagesse

montre que cette proposition de loi ne pouvait pas être votée conforme. Il a fallu auditionner un certain nombre de praticiens, notamment des notaires de Saint-Martin, pour s'en rendre compte.

ou au moins un indivisaire établi à l'étranger. La mise en place de délais différents selon le nombre et le lieu de domiciliation des indivisaires complexifierait excessivement le dispositif. On pourrait, la perspective d'une évolution du présent texte, réfléchir plutôt à un dispositif s'apparentant au « délai de distance » prévu dans le code de procédure civile. Je n'ai malheureusement pas eu suffisamment de temps pour examiner cette possibilité, mais

courant à compter de la signification du projet de vente ou de partage qui leur est faite, et ce d'autant plus que l'opposition est faite sans forme. Ainsi, un simple courrier adressé au notaire chargé de la vente ou du partage suffit. Par ailleurs, le délai d'opposition de trois mois est déjà celui du droit commun de l'article 815-5-1 du code civil. Toutefois, je peux comprendre votre souhait de parfaire l'effectivité du droit d'opposition,

qui sera donc portée par le groupe majoritaire à l'Assemblée nationale, auquel il appartiendra de trouver le créneau adapté. Pour autant, le Gouvernement

de sagesse qu'elle a exprimé me laissent à penser que le délai de trois mois peut ne pas paraître suffisant non plus, même si elle dit le contraire. J'aurais préféré, à la limite, qu'elle me dise que

La situation à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy a ceci de spécifique que de nombreux Saint-Barths et Saint-Martinois vivent à l'étranger. J'entends bien le rapporteur quand il dit que ce sujet est formidable et que l'on pourrait poursuivre cette discussion, mais, si le Sénat ne l'a pas actée,

Ces amendements visent à étendre la procédure de cantonnement en dehors des hypothèses où il existe un testament. La procédure de cantonnement a été créée par la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, au profit des légataires ou du conjoint survivant. Elle permet au bénéficiaire d'une libéralité de décider de diminuer l'étendue de l'émolument dont il aurait pu se prévaloir en application du testament, et notamment de renoncer à une partie des droits indivis auxquels il avait droit. Cette procédure, prévue à l'article 1002-1 du code civil pour les légataires, n'est pas applicable en l'absence de testament. Les amendements n 1 et 2, qui me semblent redondants, visent à permettre l'application de ladite procédure à des successions dans lesquelles il n'y a pas de testament. Actuellement, en l'absence de testament, si un héritier indivisaire décide de renoncer à ses droits au moment du partage, cette renonciation s'apparente à une libéralité faite aux autres indivisaires, taxés en conséquence. Cette idée mérite d'être approfondie, car, comme le souligne l'auteur des amendements, cette impossibilité pour l'un des indivisaires de renoncer à sa part dans l'indivision ou au versement d'une soulte qui lui serait due est un facteur important de blocage du partage. Il me semble cependant

Le cantonnement est la limitation de l'assiette d'un droit à certains biens. Il est ainsi prévu pour l'exécution d'une libéralité à la demande du gratifié, qu'il soit légataire ou conjoint survivant. Cela lui permet de choisir, au sein des biens indivis auxquels sa libéralité lui donne vocation, ceux qu'il souhaite conserver. Ici, l'hypothèse visée est tout autre. Il s'agit du cas d'un partage en nature du bien, avec allotissement d'un ou de plusieurs indivisaires du bien contre paiement d'une soulte aux autres indivisaires. L'amendement vise à permettre à certains de ces autres indivisaires de renoncer à percevoir tout ou partie de leurs droits et de leurs parts pour éviter ou limiter les soultes. On s'éloigne ainsi, me semble-t-il, assez largement de la notion même de cantonnement. En outre, cet amendement vise tous les copartageants et donne donc l'impression de ne pas viser que les seuls partages consécutifs à une succession. La mention selon laquelle le cantonnement permet d'éviter ou de limiter les soultes n'est ici ni claire ni réellement normative et peut donc prêter à des interprétations différentes. Il me semble que vous souhaitez traiter le cas d'un bien dont l'attribution à un ou plusieurs indivisaires conduirait à mettre à leur charge une soulte excessive au regard de leurs facultés. Cette situation est réglée par la jurisprudence, qui considère de façon constante que, lorsqu'il est impossible de composer des lots d'égale valeur sans mettre à la charge de certains attributaires des soultes excessives, il y a lieu de vendre les biens de façon à répartir le prix également entre les copartageants. Doit-on encourager ces renonciations au paiement de la soulte par une disposition générale permettant d'éviter leur assimilation à une libéralité et d'écarter le paiement de droits de mutation à titre gratuit ? Le Gouvernement n'y est pas favorable. Enfin, sur le plan fiscal, en se limitant aux seuls immeubles situés en outre-mer, cet amendement s'expose, me semble-t-il, à une censure du Conseil constitutionnel pour cause de rupture d'égalité avec la généralité des redevables de droits d'enregistrement et de droits de mutation à titre gratuit qui souhaitent sortir d'une indivision. Pour ces raisons,

a opté pour une rédaction scrupuleuse, à la suite de ses échanges longs et nourris avec des spécialistes du sujet, afin que le texte proposé recueille l'adhésion de l'ensemble de la classe politique. Pour ce faire, il a logiquement écarté toute mesure hasardeuse et compliquée qui pourrait mettre à mal le vote de ce texte dans les deux assemblées, avec l'objectif d'une application rapide eu égard à l'urgence de la situation dans nos territoires. m'explique pourquoi il a été ajouté par amendement une mesure fiscale d'exonération de droit de partage. Pour rappel, ce taux de 2,5 % est appliqué lors d'une rupture d'indivision entre héritiers au cours d'une succession, ou entre époux après un divorce. De plus, à la suite d'une question d'un député qui évoquait la possibilité de réduire ce pourcentage à 1 % en cas de partage rapide- réalisé en moins d'un an -, dans le but d'inciter les particuliers à accélérer les procédures, le ministre des finances a révélé que cette taxation procurait un rendement annuel de 500 millions d'euros et que, en conséquence, il était inenvisageable de diminuer cette recette. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'intéresser à cette question et, le cas échéant, Je considère sincèrement qu'une telle mesure n'a pas lieu d'être dans un texte traitant de solutions urgentes à mettre en oeuvre face aux difficultés liées à l'immobilisation du foncier. En effet, les blocages de successions en indivision sont de plus en plus nombreux et impactent fortement l'ensemble de nos territoires ultramarins. C'est pourquoi, indépendamment du bien-fondé ou non de la mesure instituée par cet article, je voterai

L'histoire marche à l'envers : généralement, c'est nous qui faisons la loi, et ce sont eux qui sont chargés de la mettre en oeuvre. Aujourd'hui, cela a été le contraire : nous avons été sous leur dictée, hélas ! La commission des lois a adopté un amendement qui prévoit une exonération de droit de partage jusqu'en 2028 des immeubles situés dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

la mesure adoptée par la commission des lois va faire obstacle à l'adoption définitive de ce texte. Il suffit de reprendre la proposition exprimée par le Gouvernement à l'Assemblée nationale. La ministre Annick Girardin a plusieurs fois émis une fin de non-recevoir sur toute question fiscale- je crois que c'est la règle de la mandature.

à l'ensemble des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ainsi qu'aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon et de prolonger cette exonération jusqu'en 2028.

2. Une disposition de même nature a été censurée par le Conseil constitutionnel, au motif que le maintien d'un régime d'exonération applicable aux successions des immeubles situés dans une zone spécifique- au cas d'espèce en Corse -méconnaissait le principe d'égalité devant la loi et les charges publiques. Il s'agit d'une décision de 2012. En outre, il est signalé que la mesure adoptée dans la loi du 28 décembre 2017 consistant à accorder une exonération temporaire de droit aux seuls immeubles situés à Mayotte n'a pas fait l'objet d'un examen au fond par le Conseil constitutionnel. Par ailleurs, cette exonération était alors motivée par l'objectif de favoriser la constitution

est l'avis de la commission ? Les amendements n 8 et 10 visent à supprimer l'exonération de droit de partage pour les immeubles situés dans les territoires ultramarins concernés par le dispositif dérogatoire de sortie d'indivision. Cette incitation fiscale a été mise en place par la commission afin d'encourager les indivisaires à sortir de ces situations problématiques, car leur généralisation dans les territoires ultramarins aboutit à une paralysie du foncier qui n'est pas sans conséquences économiques, sanitaires et sociales. Cette dérogation au régime de droit commun est prévue pour une durée strictement nécessaire au règlement des désordres fonciers ultramarins. L'exonération, comme le dispositif de sortie d'indivision, prendrait fin le 31 décembre 2028.

est à Mme la garde des sceaux. Cet amendement vise à supprimer l'article 5 A portant sur le partage par souche en Polynésie française. Je m'en suis déjà expliquée dans mon propos introductif. Je rappelle que la souche est un mode de partage du patrimoine quand l'héritier légal est lui-même décédé, permettant que les petits-enfants succèdent à leurs grands-parents par représentation de leur père ou de leur mère prédécédés. Ces héritiers, qui viennent en représentation de leur auteur prédécédé, constituent donc une souche. Pour autant, ils ne se représentent pas entre eux et ils sont tous parties au partage de la succession. L'article 5 A, en affirmant un principe de partage par souche, manque son objectif, qui est de pouvoir permettre un partage judiciaire sans besoin d'identifier ni d'appeler tous les héritiers à la cause. Je le répète, un partage par souche n'induit aucune représentation procédurale des héritiers au sein d'une même souche et chacun des héritiers a le droit d'être appelé au partage. Permettre la réalisation d'un partage judiciaire à l'insu de l'un des intéressés est une atteinte directe au droit au recours et à l'accès aux juges, qui sont des principes dont la protection est assurée, vous le savez, tant par la Constitution française que par la convention européenne des droits de l'homme. Par ailleurs, l'article 5 n'a aménagé aucune garantie ni aucun garde-fou destiné à préserver les droits des héritiers omis du partage judiciaire, alors même que les successions sont justement un domaine dans lequel les divergences d'intérêts entre les parties sont fréquentes. Il sera relevé que le rapport sénatorial du 23 juin 2016 avait, à juste titre, insisté sur la nécessité d'établir des garde-fous pour garantir les droits des indivisaires omis et d'éviter que « l'introduction d'une présomption de représentation au sein d'une souche dispense de rechercher le plus d'indivisaires possible pour les attraire au partage, et aboutissent à des partages iniques à l'insu de certains indivisaires L'organisation d'une présomption de représentation au sein de la même souche suscite également un certain nombre de questions auxquelles il n'est apporté aucune réponse. Par exemple, comment et par qui le représentant de la souche est-il désigné ou choisi ? Quel rôle exact joue le membre de la souche choisi par le demandeur au partage pour représenter procéduralement cette souche ? Doit-il aussi être considéré comme représentant d'autres membres de la souche dans la gestion du lot revenant à celle-ci, etc. ? En l'état, vous l'aurez compris, la disposition envisagée dans la proposition de loi se heurte à de nombreuses difficultés juridiques qui rendraient son application impossible. Le Gouvernement propose donc de la supprimer. Néanmoins, comme je vous l'ai déjà dit, je souhaite que la question de l'indivision en Polynésie française et du partage par souche soit examinée sérieusement par mes services, en lien avec ceux du ministère des outre-mer. Mon cabinet a donc déjà commencé ce travail avec les élus polynésiens. Je crois nécessaire que nous allions plus loin rapidement pour mesurer clairement les enjeux juridiques et apporter des solutions concrètes aux difficultés rencontrées d'un sujet sérieux, sur lequel nous devons trouver un équilibre entre le respect des principes, comme le droit de propriété

revenir sur une disposition introduite dans le texte par la commission, sur l'initiative de notre collègue Lana Tetuanui. L'article 5 A consacre la possibilité de procéder, en Polynésie française,

tel qu'il est prévu à l'article 827 du code civil est bien souvent soit impossible, soit dénué de sens au regard de l'étroitesse des parcelles et du nombre d'héritiers. La cour d'appel de Papeete a validé le principe d'un partage par grande souche familiale, cela est possible, des demandes de partage par tête au sein de chaque souche. Cette construction prétorienne vise à admettre la représentation, dans la procédure de partage, des indivisaires, qui ne peuvent être appelés à l'instance par un parent issu de la même souche. souche. Néanmoins, l'objet de cet amendement le rappelle, la Cour de cassation invalide systématiquement tous les arrêts de la cour d'appel retenant cette solution juridique, qui élargit libéralement la notion de représentation. Cette position de la Cour de cassation, aussi juste et juridiquement rigoureuse soit-elle, entraîne de lourds préjudices et retarde le traitement de la question foncière en Polynésie. Il faut admettre qu'il n'y a bien souvent pas d'autre choix que le partage par souche, comme l'ont unanimement tous les magistrats rencontrés par la délégation sénatoriale et par les membres de la commission des lois lors de leur déplacement à Papeete et dans les archipels. D'ailleurs, malgré la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le tribunal de première instance et la cour d'appel de Papeete maintiennent leur solution prétorienne. Peu de pourvois en cassation sont constatés, bien que l'invalidation soit assurée et constitue un motif général d'insécurité des partages. L'article 5 A donne donc un fondement légal à cette construction prétorienne de la cour d'appel de Papeete. Papeete. Le dispositif est-il perfectible ? Très certainement. Est-ce une raison pour les supprimer purement et simplement, alors qu'il répond à un véritable besoin et à une demande très ancienne des magistrats en exercice en Polynésie ? Je ne le pense pas. Mettons à profit la navette pour l'améliorer, plutôt que de ne rien faire en arguant des travaux en cours

Nos histoires communes ne sauraient être étranglées par le fétichisme d'un article de la Constitution. Assemblons donc tout ce qui se ressemble. Par conséquent, c'est avec un réel plaisir que j'accède j'accède à la demande pressante de mes collègues Michel Magras et Guillaume Arnell d'insérer nos compatriotes de Saint-Barthélemy

Dans chacune des collectivités, ce travail a en effet mis en lumière à quel point cette problématique pouvait souvent constituer un noeud gordien entravant la politique d'aménagement du territoire et, plus généralement, le développement dans des territoires notamment marqués par un important besoin en logements. Mes collègues ont largement souligné les difficultés engendrées par l'indivision, je ne m'y étendrai pas. Je souhaite toutefois souligner à mon tour que, en matière d'indivision, la réalité ultramarine, malgré des traits communs, n'est, là encore, pas homogène. À Saint-Barthélemy, par exemple, la situation est beaucoup plus nuancée que dans d'autres territoires, même si, comme ailleurs, la question de l'indivision s'explique souvent par la complexité des rapports entre membres d'une même famille. J'en profite pour remercier Catherine Conconne, qui a accepté une dose de différenciation territoriale. Je souscris par

Nous ne sommes pas ici à l'Assemblée nationale, nous sommes au Sénat, je tenais à le rappeler à certains de nos collègues. Lorsque la proposition de loi est arrivée de l'Assemblée nationale, elle omettait certaines collectivités, comme Saint-Martin

les deux amendements que vous n'avez pas adoptés, parce que c'est la richesse des débats au Sénat qui a mené à cette décision finale. Personne ne